La séance est ouverte.

est adopté sous les réserves d'usage. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie hier ont été adressées par courriel et sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.-

le candidat Emmanuel Macron s'était réclamé d'un point d'équilibre entre libérer et protéger. Où en sommes-nous onze mois après son élection et dix mois après un exercice, pour le moins, pyramidal du pouvoir ? Les Français sont inquiets. Qu'ils soient fonctionnaires, retraités, cheminots, personnels soignants, acteurs du logement social, étudiants, bénévoles associatifs ou élus locaux, ces Français ne voient pas l'équilibre de l'engagement présidentiel. Ils nous le disent chaque jour depuis des semaines : le compte n'y est pas La France n'est pas une start-up où le désordre deviendrait une énergie créatrice. Notre pays a besoin d'un climat apaisé et d'un cap. Votre feu d'artifice de réformes correspond-il à ce cap ? Quelle est votre vision de la justice sociale ? Quelle est la place du service public dans vos choix politiques ? Je vous pose ces questions, parce que les Français se les posent Notre pays et les Français ne sont pas contre les réformes par principe. Ils demandent d'abord à les comprendre et, surtout, à ce qu'elles portent un progrès social. Cela a toujours été notre position, celle de la responsabilité et de la recherche de l'intérêt général. Je vous pose ces questions, parce que, entre la promesse des annonces et le contenu réel des réformes, l'écart est parfois grand- nous le verrons par exemple demain avec feu l'idée d'une assurance chômage universelle Je vous pose ces questions, parce que malgré les accusations, l'été dernier, de budget insincère et de mauvaise gestion, tout le monde voit aujourd'hui que, grâce aux cinq dernières années, votre gouvernement dispose de la meilleure situation économique et financière que la France ait connue depuis plus de dix ans.

esbaudir les Français par un tourbillon de réformes ... Je ne le crois pas. Nous essayons, sujet après sujet, de réparer un pays qui a des atouts considérables et des richesses merveilleuses, mais qui connaît aussi des problèmes dont nul ici ne peut nier l'importance et l'intensité, ni l'ancienneté. Lorsque nous essayons, comme aujourd'hui, d'apporter une réponse face à la dégradation du service public ferroviaire,

ordonnances prises au mois d'octobre dernier, nous le faisons parce que, depuis trop longtemps, nous considérions que le droit du travail n'offrait pas les souplesses permettant aux petites et moyennes entreprises de recruter sans risque.

mais rien, monsieur le président Kanner, absolument rien ne nous fera dévier de cet objectif simple et des engagements qui ont été pris devant les Français.

La réformer est une nécessité, sous peine de la voir sombrer en raison d'une dette abyssale. Depuis quatre-vingts ans, les Français contribuent à la construction, à l'entretien et à la modernisation de nos rails. Du fait de cette contribution publique au financement du rail, il me semble nécessaire que les Français aient leur mot à dire sur l'avenir de ce secteur. La seule ambition que nous devons poursuivre, c'est finalement l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers

Cet après-midi, la ministre des transports rencontre les syndicats pour évoquer avec eux les enjeux de cette réforme à venir. Or les Français contribuent aujourd'hui au financement du secteur ferroviaire par l'impôt. Mais quelle place ont-ils dans les débats sur l'avenir du rail ?

Les orientations budgétaires pour 2018 du Centre national pour le développement du sport, le CNDS, ont été récemment publiées. Elles inquiètent grandement le milieu sportif. Aujourd'hui, nombre de fédérations et de comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs rencontrent de grandes difficultés face à l'amputation de l'enveloppe territoriale de près de 40 % et en raison des nouveaux critères d'attribution de financements aux associations. Depuis un an, beaucoup de messages envoyés au mouvement sportif sont très négatifs. Le budget des sports est en baisse et celui du CNDS a été divisé par deux. Le Sénat avait pourtant adopté, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2018, un amendement qui permettait de maintenir le prélèvement sur les gains de la Française des jeux affecté au CNDS à la hauteur de celui de 2017, soit 63,8 millions d'euros supplémentaires. Comme cela était malheureusement prévisible, votre majorité « En Marche » l'a rejeté à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous ciblez les financements, vous oubliez des pans entiers du territoire, vous mettez de côté certaines pratiques et enfin vous réduisez, voire supprimez l'accompagnement financier de la formation de milliers de bénévoles. Madame la ministre, alors que vous souhaitez promouvoir la pratique sportive en France, ce gouvernement réduit de manière continue les moyens d'action de votre ministère. Il pénalise le CNDS, qui était un moyen efficace de financer le sport et les infrastructures.

Comme vous le savez, le CNDS était en péril il y a quelques années. Pour l'année 2018, il bénéficie d'un budget de 153 millions d'euros, à replacer dans le contexte d'une réduction globale des dépenses publiques que vous connaissez- je crois d'ailleurs que vous partagez

les projets des associations locales et à résorber les inégalités territoriales. L'établissement conservera une enveloppe dédiée au soutien à la création et à la rénovation d'équipements sportifs pour les territoires les plus carencés-

que l'intervention de l'État auprès des partenaires associatifs et des clubs doit répondre au devoir de sobriété et d'efficacité, en évitant le saupoudrage en matière de subventions. Monsieur Savin,

de la santé. Le nombre d'agressions de médecins vient d'atteindre un nouveau record. Selon une récente étude du conseil national de l'ordre, plus de 1 000 médecins ont été agressés en 2017. Ce nombre a considérablement augmenté depuis 2003. Les praticiens les plus visés sont les généralistes et les femmes, majoritairement en milieu urbain. Ces chiffres sous-estiment sans doute la réalité, car il est évident que toutes les agressions ne sont pas répertoriées, faute d'un dépôt de plainte systématique par les victimes. Comme de nombreuses autres professions, les médecins sont confrontés chaque jour à des personnes qui perdent leurs moyens face à des situations de détresse. Ils savent alors faire preuve de pédagogie, rassurer et apaiser. La plupart du temps, la tension retombe. J'ajoute que les dysfonctionnements de notre système de santé les exposent encore plus, car, pour les patients, à l'angoisse de devoir lutter contre la maladie s'ajoute celle de devoir s'orienter dans un environnement complexe. Mais il y a des situations que les médecins ne peuvent ni éviter ni anticiper : cela va des incivilités quotidiennes aux agressions physiques- crachats, coups ... -, voire aux agressions sexuelles. En ville ou à l'hôpital, la médecine est une vocation pour celles et ceux qui l'exercent. Ils doivent déjà, quotidiennement, surmonter de nombreux obstacles. Partout, le point de rupture est atteint, ou près de l'être. Au manque de moyens et de reconnaissance s'ajoute l'insécurité : même les vocations les plus affirmées n'y résisteront pas longtemps. Comment avons-nous pu laisser ce climat de violence s'installer ? Comment avons-nous pu laisser cette violence prospérer d'année en année sans rien faire, ou presque ? Madame la ministre, face à cette situation intolérable, quelles mesures votre gouvernement compte-t-il mettre en oeuvre pour protéger nos médecins ?

La politique de prévention et de lutte contre les violences est un axe majeur développé par le ministère des solidarités et de la santé, tant à l'égard des établissements de santé qu'au profit de l'ensemble des professionnels. L'Observatoire national des violences en milieu de santé signale chaque année les agressions qui ont lieu dans les établissements de santé

où vous avez eu l'occasion de rencontrer le président de la République d'Arménie, M. Serge Sarkissian, et de participer à des échanges sur les moyens de renforcer la coopération et nos liens économiques, politiques et culturels avec ce pays ami de la France.

l'écrin de toutes les autres et nous n'avons de cesse de la partager avec tous ceux qui la parlent. Dans son discours à l'Institut de France, le Président de la République a parlé, je le cite, de ces valeurs qui nous guident et qui doivent également guider notre action en matière internationale.

dans ce domaine d'ici octobre prochain, notamment celles qui concernent la promotion culturelle et politique du français à l'étranger, au-delà des traditionnels pays dits francophones. La parole

collègues, ce lundi 2 avril avait lieu la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À cette occasion, le Gouvernement a annoncé vouloir mettre l'accent sur le diagnostic dans le cadre du quatrième plan Autisme. En matière de diagnostic chez l'enfant, la France a fait beaucoup de chemin ces dernières années, mais on estime encore que seulement 10 % des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme sont aujourd'hui diagnostiquées. Des efforts considérables restent donc à faire, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. J'aimerais, pour ma part, vous interroger sur la place accordée, dans ce nouveau plan, à une recommandation de la Haute Autorité de santé. Dans son avis rendu public le 19 février dernier, la HAS insiste sur l'importance d'associer les personnes autistes et leurs familles, à chaque étape de leur parcours, à la prise de décision et à la définition de leur projet personnalisé. L'objectif est, bien sûr, le respect des droits des personnes, mais aussi une meilleure coordination entre leurs volontés, leurs capacités et la place que la société peut leur offrir. Car chaque personne est différente et l'on ne peut se satisfaire d'une solution appliquée à tous. Le virage inclusif a permis d'ouvrir l'école aux enfants autistes et le monde du travail aux adultes. Il a également permis de démontrer que, en considérant chaque différence comme une chance, c'est la société dans son ensemble qui était gagnante. Mais, puisque l'étendue du spectre est immense, les solutions proposées doivent l'être aussi. Certains s'épanouissent en structure d'accueil spécialisée, tandis que d'autres travaillent en milieu ordinaire et font preuve de compétences que nous, neurotypiques, ne serons jamais en mesure d'acquérir. Dans tous les cas, même lorsque les difficultés de communication sont un frein, nous devons être en mesure de comprendre et d'appréhender les besoins de chacun. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous détailler les mesures prévues par le Gouvernement pour un plus grand respect des droits et des choix des personnes autistes ? La parole

directement ou indirectement par l'autisme nous disent combien il est important que les alertes données par les parents soient prises au sérieux le plus en amont possible, afin que l'on puisse apporter la réponse la plus efficace et la plus personnalisée.

d'abord de donner enfin une place aux personnes autistes dans la cité. Vous l'avez dit, des progrès ont été réalisés à cet égard, mais d'autres doivent encore l'être, notamment à l'école, dans le monde du travail, dans les activités sociales et culturelles, en transformant en profondeur la manière de travailler des services, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, afin qu'ils interviennent au bon moment, au bon endroit, auprès de la bonne personne. Vous le voyez, le Gouvernement est pleinement mobilisé. Le Président de la République a profité de son déplacement aujourd'hui à Rouen

Le Président de la République a fait une erreur qu'il risque de payer, celle de tenter de diviser notre peuple, en opposant, par exemple, les retraités agricoles aux cheminots. Il a fait une erreur en traitant de privilégiés ceux qui travaillent dur et de délinquants potentiels ceux qui ne travaillent pas. L'impact de ces erreurs et de ces provocations est démultiplié par l'affichage d'une présidence pour les riches, avec l'hallucinante suppression de l'ISF pour les actionnaires, qui fournissent pourtant le gros des bataillons des évadés fiscaux ! Le Président de la République a fait une erreur, car il a profondément sous-estimé l'attachement de notre peuple au service public, à l'intérêt général, à l'égalité. La lutte des cheminots, monsieur le Premier ministre, est comprise d'une large majorité d'usagers qui connaissent eux aussi, dans leur entreprise, chez Carrefour par exemple, la violence sociale. Toutes et tous ont besoin du service public que vous menacez ! La mobilisation des étudiants contre Parcoursup et la ségrégation sociale vous surprend. Vous pensiez avoir réglé la question par un débat express au Parlement et une application précipitée des nouvelles règles de sélection. Là aussi, c'était sans compter sur l'attachement profond de notre jeunesse à l'égalité et à l'intérêt général. Cette mobilisation rejoint celle des retraités, des fonctionnaires, du monde de la justice, du secteur de la santé, ainsi que la lutte des cheminots. vous devez prendre conscience de la colère qui monte contre cette politique. Vous devez stopper cette avalanche de projets et de mesures imposés sans débat ou presque. Monsieur le premier ministre, allez-vous faire le choix de l'affrontement social ?

généralisée. Nul ici ne pourra le contester, j'ai toujours marqué le plus grand respect pour les libertés constitutionnellement garanties, dont la liberté de faire grève.

Notre objectif, madame Assassi, est non pas de casser le service public, comme vous l'affirmez parfois, mais, au contraire, de faire en sorte que, dans le monde

Gouvernement. La santé est une responsabilité de l'État. Or, depuis l'incendie du CHU de Pointe-à-Pitre, le 28 novembre dernier, la Guadeloupe connaît une situation d'urgence sanitaire sans précédent.

mes questions relaieront les attentes légitimes des Guadeloupéens. Pouvez-vous, devant la représentation nationale, rétablir la vérité sur la sécurité sanitaire en Guadeloupe et enfin redonner confiance aux usagers et au personnel ?

Guadeloupe, l'établissement a dû être totalement évacué. Le CHU a été réinvesti progressivement à partir du 7 janvier dernier, après un nettoyage en surface des locaux. Cette réintégration a permis de répondre sur place et rapidement aux besoins sanitaires de la population. Sur les 563 lits disponibles en 2017, 418 étaient réinstallés au 16 mars 2018, au CHU, mais également chez ses partenaires : la clinique des Eaux-Claires, la clinique de Choisy, la polyclinique de Guadeloupe et le centre hospitalier de Basse-Terre. Des expertises techniques ont été diligentées concernant, d'une part, la santé des patients et du personnel, et, d'autre part, le bâtiment et les risques éventuels encourus. L'absence de risque grave et imminent pour les personnes a été soulignée par les opérateurs. Il est cependant apparu indispensable, pour l'exploitation sur le long terme de l'hôpital, de réaliser un nettoyage méthodique en profondeur. Suivant les conseils des experts, le nettoyage de la tour nord doit être effectué en site totalement vide. Les différents services seront donc réorganisés en lien avec les établissements partenaires et un pôle mère-enfant sera constitué à la polyclinique de Guadeloupe. Les modalités du nettoyage du plateau technique et de la tour sud sont, quant à elles,

sur plusieurs mois, selon un phasage précis, qui nécessitera un confinement très rigoureux et maîtrisé des locaux. En revanche, si les travaux ne peuvent être réalisés en site occupé, la mise

dès le démarrage du traitement ou sa suppléance. Il faut également améliorer l'information sur les modalités de traitement existantes, ainsi que l'éducation thérapeutique. Enfin, il convient de renforcer la prise en charge en amont. Tout cela devrait permettre, monsieur le sénateur, de limiter ou de retarder

Tout exploitant d'un établissement comportant un débit de boissons à consommer sur place qui souhaite accueillir un mineur de moins de seize ans, qu'il s'agisse d'un élève d'un lycée professionnel, d'un apprenti ou d'un salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation, doit obtenir au préalable un agrément. Cet agrément constitue une dérogation au principe selon lequel il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Vous n'êtes cependant pas sans savoir, monsieur le ministre, que les jeunes sortant de troisième aujourd'hui, et donc éligibles à l'apprentissage ou aux stages, ont, du fait d'un faible taux de redoublement, moins de seize ans, voire moins de quinze ans. On peut s'en féliciter,

opposer une fin de non-recevoir. Pour étayer mon propos, je prendrai l'exemple concret d'une région que je connais bien, le Grand Est, où quelque 300 jeunes qui auraient souhaité apprendre les métiers du service en restauration à la rentrée prochaine se trouvent complètement démunis. À l'heure où le Gouvernement entend faire du développement de l'apprentissage une de ses priorités, comme en témoigne le projet de loi de réforme de l'apprentissage que nous aurons l'occasion d'examiner prochainement,

Comment comptez-vous, monsieur le ministre, remédier à cette difficulté pratique, sachant qu'il y a urgence à agir, puisque la rentrée des futurs apprenants se prépare dès maintenant ? Pouvons-nous compter sur vous dans la perspective de l'examen du projet de loi que je viens de mentionner ?

Merci,

les collectivités territoriales sont tenues de participer, sous forme de l'acquittement d'un forfait, au fonctionnement matériel des écoles, des collèges et des lycées sous contrat d'association avec l'État. Cette obligation vaut aujourd'hui uniquement pour les élèves pris en charge à partir de l'âge de six ans, auquel la scolarité devient obligatoire. Le Président de la République a affirmé le 27 mars dernier, en ouverture des Assises de l'école maternelle, sa volonté d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire à trois ans. Nous sommes nombreux, au sein de cet hémicycle, à nous féliciter de cette décision sur un plan éducatif. Toutefois, nous nourrissons d'importantes inquiétudes quant à ses conséquences financières, qui pourraient être beaucoup plus lourdes pour nos communes que pour l'État. En effet, à ce jour, les enseignants des écoles maternelles privées sous contrat sont déjà rémunérés par l'État. En revanche, la participation des communes, dans le cadre du forfait d'externat, n'est pas légalement requise. Mais si l'âge de la scolarité obligatoire était abaissé à trois ans, les écoles maternelles privées sous contrat seraient en droit de réclamer une contribution aux communes qui n'en apportent pas déjà une sur la base du volontariat. En outre, le forfait couvrant les frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat étant indexé sur les dépenses des communes pour l'école publique, nous savons qu'il sera plus élevé pour les écoles maternelles, du fait notamment de la présence des ATSEM,

Par une circulaire du 12 décembre dernier, M. le ministre de l'intérieur a chargé les préfets d'organiser le contrôle des centres d'hébergement d'urgence pour y collecter des informations sur la situation administrative des personnes qu'ils accueillent, cela en vue d'éviter la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence. Il me paraît en effet naturel, même si cela peut choquer certains, que l'État puisse s'assurer des conditions de séjour des personnes accueillies dans des centres financés par de l'argent public. Aujourd'hui, il semblerait que certaines des 140 000 personnes hébergées ne devraient plus l'être ou soient sans statut, ce qui ne permet plus d'accueillir de potentiels nouveaux bénéficiaires. L'objet de cette circulaire me paraissait donc parfaitement légitime. Pourtant, sur le terrain, la pratique est très éloignée de la communication, dans la mesure où les équipes dans la mesure où les équipes mobiles chargées de cette mission ne peuvent recueillir des informations sur les personnes hébergées que si ces dernières Je souhaiterais donc savoir combien d'équipes mobiles ont été réellement créées et combien de centres d'hébergement ont été effectivement contrôlés depuis la publication de cette circulaire. Comment les personnes identifiées comme ne devant plus être hébergées dans ces établissements ont-elles été concrètement prises en charge et réorientées ? Pour le groupe Les Républicains comme, me semble-t-il, pour beaucoup de Français, l'exercice du droit à l'hébergement d'urgence n'exclut pas le respect des devoirs qui y sont liés.

Vous l'avez rappelé, des équipes mobiles composées d'agents de préfectures et d'agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été chargées d'examiner la situation administrative des personnes accueillies dans les centres d'hébergement d'urgence, ainsi que

L'objectif est donc d'abord de connaître la situation des personnes afin de leur proposer au plus vite une solution adaptée. Vous m'avez posé des questions très précises,

-une décision prise au mépris du plan de déplacements urbains d'Île-de-France, dont le périmètre a été fixé à l'échelon du territoire régional. Est-il besoin de rappeler ici que cette décision a été prise malgré l'avis défavorable de la commission d'enquête et l'opposition de la majorité des riverains ? Aujourd'hui, à l'heure où le débat sur le périmètre exact du Grand Paris fait rage, ce triste épisode de la fermeture des voies sur berges apporte la preuve concrète que c'est bien la région qui fait métropole. En effet, les Franciliens sont tous concernés par cette décision aveugle et dogmatique. Pour eux, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Autour de la capitale, les temps de trajet ont bondi. Ainsi, les habitants de l'Essonne, territoire

La qualité de l'air s'est-elle améliorée ? Non ! Le bruit a-t-il diminué ? Merci, chers collègues ! Monsieur le ministre, nous défendons, dans cet hémicycle, le principe de réalité. Nous plaidons pour le droit à l'expérimentation selon une formule simple et pragmatique : ce qui fonctionne doit être conservé, ce qui ne fonctionne pas doit être abandonné il est grand temps de rouvrir les voies sur berges à la circulation et d'engager une véritable concertation au niveau régional ! Pour sa part, la présidente de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, y est prête. Elle a même déjà fait des propositions concrètes. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que soit respecté le plan de déplacements urbains d'Île-de-France et que cesse enfin ce qui est devenu un véritable problème d'ordre public ?

demande du groupe du RDSE, de la proposition de loi relative à l'élection des conseillers métropolitains, présentée par Mme Mireille Jouve et plusieurs de ses collègues

feront l'objet, lors de leur prochain renouvellement, d'une élection au suffrage universel direct selon des modalités fixées par une loi promulguée avant le 1 janvier 2019. 2019. S'il n'entraîne aucune obligation à l'égard du législateur, l'article est de nature à créer une incertitude parmi les élus locaux concernés. Sa suppression aurait indéniablement le mérite d'apporter de la clarté, de la stabilité et de rappeler l'attachement du Sénat

des métropoles. À l'exception du Grand Lyon, toutes les métropoles françaises demeurent, à ce jour, des établissements publics de coopération intercommunale. Admettre une élection au suffrage universel direct des conseils métropolitains dans le cadre d'un scrutin distinct reviendrait inexorablement à séparer communes et métropoles et à transformer ces dernières en collectivités territoriales. Or l'intercommunalité a été pensée et conçue comme une émanation des communes dont la vocation première est la mutualisation des compétences et la création d'une gouvernance de projets. Elle repose aussi sur le principe de subsidiarité. À cet égard, que restera-t-il aux communes métropolitaines, une fois qu'elles auront transféré leurs compétences, coopéré de bonne foi à la gouvernance avant de voir le lien qui les unit à la métropole définitivement coupé, et cela, cruel paradoxe, alors que les élus municipaux continueront d'être interpellés par leurs administrés ? La mort annoncée de ces communes, nous la refusons L'échelon communal demeure, j'en suis convaincue, la clef de voûte de la cathédrale républicaine. Je reconnais volontiers, mes chers collègues, que les détracteurs les plus assidus du socle communal ne siègent pas au sein de cet hémicycle, mais la rengaine, hors de ces murs, est souvent la même.

La France comptait 38 000 communes en 1789. Elles sont environ 35 000 aujourd'hui. Depuis plus de deux siècles, la République semble s'en être accommodée. Ce qui peut apparaître à certains comme une tare ineffaçable est aussi une force, celle de la proximité, celle du lien politique et social qui unit les Français à leur maire et à leurs élus municipaux. Par les temps qui courent, cette relation est plus que jamais précieuse pour maintenir notre cohésion nationale. Nous comprenons les attentes qui peuvent conduire certains présidents d'exécutifs métropolitains à réclamer un scrutin distinct de celui des communes, et donc détaché Comme avait coutume de dire Clemenceau, « pour prendre une décision, il faut être un nombre impair de personnes, et trois, c'est déjà trop ». Nous entendons également les motivations de celles et de ceux qui, membres de formations politiques au faible ancrage territorial, voient dans l'avènement d'un scrutin de liste distinct l'occasion de s'ouvrir plus largement la porte des hémicycles métropolitains. Il nous semble cependant que le maire, parce qu'il est le maire, doit être partie prenante à la vie des métropoles. Il est et demeure, avec l'ensemble du conseil municipal, le principal interlocuteur des habitants. Il est celui qui résiste aujourd'hui le mieux à la perte croissante de crédit de la chose publique. Il est clairement identifié par le plus grand nombre.

Elle est, sur le terrain, l'oeuvre du temps, le fruit de rencontres et d'échanges multiples. Il ne nous apparaît pas faire preuve de conservatisme en rappelant ces fondamentaux ; tout au plus de pragmatisme. Si le pouvoir est lointain, inaccessible, déconnecté, alors nous gouvernerons sans les Français, et ces derniers s'éloigneront toujours davantage des urnes ... Le système du fléchage pour les communes de plus de 1 000 habitants est une création sénatoriale dont nous pouvons nous enorgueillir. Il faut le répéter, le fléchage représente bien une élection au suffrage universel direct, comme l'a reconnu le Conseil constitutionnel. Il n'est donc pas moins légitime que les trois présentés en janvier 2017, qui ont mis à rude épreuve les capacités créatives, pourtant grandes, de la Il est un second grief parfois formulé à l'encontre du fléchage : un manque de lisibilité, du fait d'une double désignation. Son intelligibilité pour le citoyen ne souffre pourtant d'aucun reproche. Elle pourrait même apparaître comme exemplaire au regard des alternatives susceptibles de lui être opposées. Je pense notamment à celle qui semblait avoir la préférence du précédent exécutif et qui s'apparentait, peu ou prou, au système en vigueur pour l'élection des conseillers régionaux. Au sein de la métropole du Grand Paris, sa mise en oeuvre aurait conduit à présenter des listes comptant au moins 209 candidats répartis dans 131 circonscriptions communales ... En termes de lisibilité du bulletin de vote, vous reconnaîtrez, mes chers collègues, que l'on a vu plus limpide Enfin- et c'est là sans doute le principal argument de celles et de ceux qui réfutent notre démarche -, le fléchage ne permettrait pas la nécessaire appropriation par nos concitoyens du fait métropolitain. Encore une fois, le système de désignation actuel ne nous paraît pas constituer un obstacle à la mobilisation des citoyens autour d'un débat et de projets métropolitains. À l'occasion des dernières élections municipales, et alors qu'il n'existait qu'une métropole, de Nice, la thématique métropolitaine avait souvent été éludée, car elle était essentiellement évoquée à propos de l'opportunité de créer, ou pas, des métropoles. Nous ne pouvons donc nous référer à aucun précédent susceptible de démontrer cette insuffisance. Or, depuis, le fait métropolitain a totalement imprégné la vie municipale dans les communes concernées. Soyez assurés que, lors des campagnes de 2020, projets municipaux et métropolitains seront au coeur des débats. Ancienne Ancienne maire sans étiquette d'une commune de 4 000 habitants, je souhaite, pour conclure, insister sur la dérive politique politique et partisane qui découlerait d'une désignation des conseillers métropolitains par le biais d'une élection autonome. Certains estiment que le système actuel ne permet pas de dégager une majorité politique claire au sein des assemblées délibérantes. Je vois pour ma part dans les hémicycles intercommunaux ou métropolitains de véritables instances de dialogue et de consensus. Dans mon département, au sein de la métropole Aix-Marseille Provence, de nombreux maires sans étiquette ne seraient plus en mesure de se situer, ou même d'exister, au sein d'hémicycles fortement « politisés », comme le sont par exemple, aujourd'hui, nos conseils régionaux.

ne plus imposer par le haut », « écouter les élus locaux » ... Les élus locaux seront tellement bien écoutés qu'ils seront purement et simplement évincés, et ce- c'est une première -à l'échelle de tout un département La précédente métropole avait peut-être été imposée par le haut, mais elle avait du moins intégré en son sein celles et ceux qui ont fait jusqu'ici la vie des territoires, désormais largement administrés par la métropole. Là encore, l'« ancien monde » est prié de faire place nette. Au-delà des seules métropoles, et pour revenir à des considérations moins provençales, je veux dire un mot de l'ensemble des intercommunalités. Lors de l'examen du projet de loi NOTRe, une disposition adoptée par les députés prévoyait l'élection de tous les exécutifs des EPCI par le biais d'un scrutin direct distinct de l'élection municipale. Si certains d'entre nous sont aujourd'hui enclins à voir dans l'article 54 de la loi MAPTAM un véritable galop d'essai, on reconnaîtra qu'il n'y a pas nécessairement lieu de les accuser de verser dans le complotisme Mes chers collègues, les signataires de cette proposition de loi ne croient pas à un prétendu « sens de l'histoire ». À cette conception hégélienne, nous opposons la phrase de Valéry : « L'histoire justifie ce que l'on veut. nous nous situons plutôt à la croisée des chemins : nous devons construire, avec les élus, un modèle d'organisation territoriale pertinent et démocratique. Les métropoles sont appelées à exercer des compétences très largement communales. Nous y souscrivons pleinement.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, bien que récentes, les métropoles créées par vagues successives suscitent des questions, parfois d'ordre identitaire, voire existentielles, grandes leurs difficultés à trouver leur place dans l'architecture institutionnelle de la décentralisation. La proposition de loi de notre collègue Mireille Jouve et de plusieurs membres du groupe du RDSE vise

Une proposition de loi identique a été déposée par notre collègue Sophie Joissains. Force est de constater que ces propositions de loi sont pleines de bon sens et de sagesse.

Les métropoles constituent aujourd'hui des objets mal identifiés, qui nécessitent selon nous une véritable évaluation. Initialement, leur création avait pour objet de permettre à quelques grandes agglomérations urbaines de renforcer leur attractivité et leur dynamisme économique dans un réseau d'échanges à vocation européenne, voire internationale. Cette dimension première ne devait concerner que quelques grandes aires urbaines. Elle a rapidement été dépassée, au bénéfice d'intercommunalités de projet,

-, de leur statut, puisque la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à part entière au sens de l'article 72 de la Constitution, tandis que les autres sont des EPCI à fiscalité propre, dont deux à statut particulier, la métropole du Grand Paris et celle d'Aix-Marseille Provence. assouplissements successifs des critères de création d'une métropole ont fortement altéré le concept. Un premier bilan de cette métropolisation accélérée est nécessaire. La mission de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre des lois de réforme territoriale installée par la commission des des lois pourrait s'atteler à ce travail, sous l'égide de son rapporteur, notre collègue Mathieu Darnaud. Concernant l'élection des conseillers métropolitains, la proposition de loi soumise à notre examen nous invite raisonnablement au. L'ambiguïté de l'article 54 de la loi MAPTAM, l'absence d'alternative crédible et notre volonté de réaffirmer la place centrale de la commune nous conduisent à soutenir clairement l'initiative du du RDSE. L'article 54 de la loi MAPTAM est en effet le fruit d'un compromis arraché en commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale étant favorable à l'élection directe des conseillers métropolitains et le Sénat y étant fortement opposé. Il comporte une clause de revoyure ambiguë et prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement avant le 30 juin 2015. Ce rapport a finalement été rendu au mois de janvier 2017. L'ambiguïté porte tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, car l'obligation de légiférer avant le 1 janvier 2019 n'engage que le législateur. Au Gouvernement ne s'impose que le respect de la tradition républicaine, qui veut que l'on ne modifie pas un mode de scrutin dans l'année qui précède l'élection concernée. Pour les élections municipales et communautaires, la date butoir est donc fixée Sur le fond, car l'article 54 de la loi MAPTAM prévoit le recours au suffrage universel direct, mais n'en précise pas les modalités. Hormis la métropole de Lyon, où la désignation directe des conseillers métropolitains est liée au statut de collectivité territoriale, les autres métropoles recourent au suffrage universel direct le mode de scrutin dit du « fléchage » pour les communes de plus de 1 000 habitants. Lors de l'examen du projet de loi NOTRe, le constat semblait largement partagé par Mme la ministre, alors sénatrice du Loir-et-Cher, qui précisait que « les élus communautaires sont d'ores et déjà élus au suffrage universel direct par fléchage ». Pour les communes de moins de 1 000 habitants, la désignation des conseillers métropolitains se fait selon l'ordre du tableau. Aujourd'hui, 96 % des conseillers métropolitains sont élus suivant le principe du fléchage sur les listes municipales, selon les règles de représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Au moment du vote, l'électeur est en mesure d'identifier les candidats aux fonctions municipales et les candidats aux fonctions métropolitaines. Il s'agit donc bien d'une élection au suffrage universel direct. L'absence d'alternative crédible est soulevée dans le rapport remis par le Gouvernement au mois de janvier 2017. Relevant qu'il n'existe aucun consensus au sein même des métropoles, ce rapport analyse trois distincts alternatifs au scrutin existant. Le premier repose sur l'existence de deux collèges, l'un composé des représentants des communes, l'autre de conseillers métropolitains élus directement. Le deuxième conçoit l'élection de l'assemblée métropolitaine dans des circonscriptions communales,

Devant l'absence de solutions alternatives crédibles, il convient donc de maintenir le système actuel. Nous rejoignons ainsi notre collègue Jean-Pierre Sueur, qui, au moment du vote de l'article 54 de la loi MAPTAM, avait précisé que « la loi fixera les modalités des élections de 2020, qui pourront être les mêmes qu'aujourd'hui Cette solution présente à mes yeux trois avantages majeurs. Premièrement, elle évite de transformer les métropoles en collectivités territoriales siphonnant les départements et les communes et complexifiant encore l'organisation territoriale. Deuxièmement, le assure la stabilité dont les collectivités territoriales ont bien besoin et la pause dans les réformes institutionnelles réclamée par de nombreux élus locaux. Enfin et surtout, le mode de scrutin actuel garantit, tout en ayant recours au suffrage universel direct, que les conseils métropolitains restent l'émanation des conseils municipaux. Le lien entre la commune et la métropole est essentiel au bon fonctionnement de l'intercommunalité.

proposition de loi vise à revenir sur le régime électoral applicable à l'ensemble que forment les métropoles au sein de la catégorie des intercommunalités à fiscalité propre. propre. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte tend non pas à faire évoluer ou à compléter les règles électorales applicables aux intercommunalités à fiscalité propre qui ont le statut de métropole, mais à les stabiliser. Permettez-moi, monsieur le président de la commission des lois, de saluer le travail réalisé en commission, qui a permis que soit examiné aujourd'hui un texte épuré, aux ambitions claires et précises. Merci ! Je concentrerai mon propos sur trois éléments qui fondent la position du Gouvernement sur cette proposition de loi.

de mars 2014, pour la première fois, nos concitoyens ont pu voter pour la désignation des conseillers communautaires, en même temps qu'ils élisaient les conseillers municipaux. C'était déjà « en même temps Cette évolution était devenue indispensable. En effet, l'extension progressive des compétences des intercommunalités, leur rôle accru dans l'organisation des des services publics locaux, mais aussi le fait que des leviers fiscaux soient à leur disposition, ont conféré aux intercommunalités une responsabilité politique croissante, que nul ne songerait aujourd'hui à remettre en cause. Toutefois, cette évolution fondamentale de l'organisation décentralisée de notre République ne s'était pas accompagnée d'une évolution des modalités de désignation des conseillers communautaires. leur légitimité était réelle, car procédant des conseils municipaux, mais elle était sans lien avec le corps électoral, avec l'expression politique et le suffrage de nos concitoyens. Cette situation nourrissait d'ailleurs des critiques récurrentes à l'égard des intercommunalités, dont le « déficit démocratique » était régulièrement dénoncé.

Dans le même temps, cette loi a permis de progresser dans la mise en oeuvre du principe de parité. Elle a constitué une avancée très importante sur ce point. sur ce point. Deuxièmement, s'agissant des métropoles, la question de la poursuite du renforcement du lien entre élus et corps électoral a légitimement été posée par le législateur. La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoyait que le Gouvernement dépose un projet de loi organisant l'élection des conseillers métropolitains

Il est vrai que l'intégration souvent plus aboutie et la dynamique récente de prise de compétences départementales des métropoles, par le biais du mécanisme de transfert prévu par la loi NOTRe, posent avec d'autant plus d'acuité la question de la légitimité démocratique des organes délibérants des métropoles. Telle est la raison pour laquelle bon nombre de ces collectivités admettent que la question de l'élection au suffrage universel direct doit être étudiée. Les travaux préparatoires aux lois MAPTAM et NOTRe l'ont amplement démontré ; certains ici s'en souviennent. ; certains ici s'en souviennent. Pour autant, à l'exception de la métropole de Lyon, qui a la qualité de collectivité à statut particulier, les métropoles se sont jusqu'à présent inscrites dans le registre de l'intercommunalité, ce qui entraîne une configuration de contraintes particulière en matière électorale. En effet, l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct sans fléchage, qu'envisageait la loi MAPTAM, est soumise à deux contraintes. part, conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la répartition des sièges au sein du conseil métropolitain doit s'opérer « sur des bases essentiellement démographiques afin de garantir l'égalité de représentativité des conseillers communautaires. D'autre part, dans le cadre de l'intercommunalité, pour assurer l'absence de tutelle d'une collectivité sur une autre, chaque commune membre de l'EPCI doit être représentée au sein de l'assemblée délibérante.

conduit nécessairement à en affecter un plus grand nombre aux communes les plus importantes, afin d'assurer l'égale représentation démographique. S'agissant des métropoles, il en résulterait des augmentations des effectifs des organes délibérants d'autant plus élevées que l'hétérogénéité démographique des communes membres de la métropole est importante. Ainsi, le rapport entre la commune la moins peuplée et la commune la plus peuplée est de 1 à 1894 à Toulouse, de 1 à 2028 à Grenoble, de 1 à 3423 à Nice,

la mise en place du suffrage universel direct sans fléchage dans le cadre de l'intercommunalité à fiscalité propre ne peut s'envisager dans le respect des principes constitutionnels sans une augmentation démesurée de la taille des conseils métropolitains ou une complexification à l'excès des modes de scrutin. Telles sont les raisons qui ont vraisemblablement conduit le précédent gouvernement à ne pas donner suite

Dès lors qu'une métropole accède au statut de collectivité à statut particulier, la configuration de règles et objectifs à valeur constitutionnelle est transformée. Les règles et principes qui caractérisent l'intercommunalité à fiscalité propre ne s'appliquent plus, puisqu'il est alors question de collectivités de plein exercice, qui s'administrent librement, par un conseil élu. élu. Par conséquent, des dispositions législatives qui organiseraient le changement de statut de certaines métropoles auraient à traiter du régime électoral qui leur serait applicable.

Sous cet angle, qui n'est plus celui de l'intercommunalité à fiscalité propre classique et qui suppose une évolution institutionnelle substantielle, la question de l'élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains pourra de nouveau être débattue devant le Parlement.

À l'issue de cette phase de réflexion, dans les conditions évoquées par le Président de la République, nous pourrons être amenés à proposer ensemble les évolutions institutionnelles, d'une part, et celles du régime électoral, d'autre part, qui trouveraient à s'appliquer à un certain nombre de métropoles. comme je vous l'indiquais, l'évolution du mode de scrutin est intimement liée aux évolutions institutionnelles. Bien évidemment, l'accès d'une métropole à la qualité de collectivité à statut particulier, collectivité de plein exercice, transforme fondamentalement les termes de l'équation du mode de scrutin. Le Gouvernement entend donc traiter ensemble de ces deux questions lorsqu'elles se poseront. Mesdames, messieurs les sénateurs, pour conclure, je vous indique que, dans le cadre de la réflexion engagée, la question du rôle et de la place des maires dans les métropoles est elle aussi bien identifiée, identifiée, tout particulièrement par le ministre d'État et par moi-même. Cette question fait partie du programme de travail du Gouvernement et pourra, elle aussi, justifier des évolutions législatives. Dans les métropoles comme dans les autres intercommunalités à fiscalité propre, chacun connaît et mesure en effet le rôle des maires dans la construction des projets communautaires.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, au sein de la loi MAPTAM a été logée une bombe à retardement son article 54, qui renvoie prudemment à une prochaine loi le soin de fixer les modalités de l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. Il s'agit d'une bombe à retardement car, mine de rien, découpler l'élection des conseillers métropolitains et celle des conseillers municipaux change la nature des intercommunalités. cessent alors d'être un outil des communes qui les gouvernaient en y envoyant des représentants élus directement par les citoyens à l'occasion des élections municipales et deviennent des collectivités autonomes

écarte l'actuel mode d'élection des représentants des communes au conseil métropolitain, au motif qu'il ne fait pas suffisamment apparaître les enjeux métropolitains et ne garantit pas qu'une majorité claire se dégage toujours au sein du conseil métropolitain ; par ailleurs, il envisage trois modes de scrutin alternatifs possibles. Outre que l'on ne connaît pas d'exemple d'intercommunalités dysfonctionnant du fait du mode d'élection des conseillers communautaires, ce qui rend ces propositions fondamentalement inacceptables, c'est que toutes changent la nature des métropoles qui, exception faite de la métropole lyonnaise, sont aujourd'hui des EPCI, des collectivités territoriales. Elles deviendraient des entités spécifiques, de véritables collectivités territoriales. Or ce qui fait l'EPCI, c'est que son conseil exprime les volontés des communes membres, ce que seuls peuvent faire des représentants de celles-ci. Contrairement à ce que laisse croire le rapport, élire des conseillers au sein d'une circonscription communale, comme le prévoient certains modes de scrutin, ne suffit pas à en faire des représentants des communes : là est l'escroquerie intellectuelle. Le mode de scrutin par fléchage ne rend pas les métropoles et ses enjeux suffisamment visibles, nous dit-on. Sauf élection dans le cadre métropolitain, les modes de scrutin alternatifs ne le permettent pas Au contraire, le mode de scrutin actuel lie les enjeux communaux et les enjeux métropolitains et place ces derniers au coeur du débat des élections municipales, qui restent les élections les plus mobilisatrices. Changer ce mode de scrutin serait clairement une étape supplémentaire du projet en cours de mise en oeuvre de dissolution des communes dans des intercommunalités qui se substitueraient à elles par siphonnage de leurs compétences et de leurs ressources. On commencera par le mode d'élection des conseillers métropolitains et l'on continuera, n'en doutez pas, par celui des conseillers d'agglomération, puis des communautés de communes importantes. Il n'en manque pas Qu'on le veuille ou non, l'actuel mode de scrutin pour l'élection des conseillers communautaires et métropolitains est le seul qui permette la représentation des communes, même les plus petites, en tant que communes, tout en respectant la règle de représentation essentiellement démographique. La proposition de supprimer l'article 54 de la loi MAPTAM doit donc être soutenue sans hésitation, d'autant que le mode de scrutin actuel permet déjà l'élection au suffrage direct de 96 % des conseillers communautaires, ceux qui sont issus des communes de plus de 1 000 habitants.

améliorer le dispositif en accordant plus de place et de moyens d'expression aux oppositions, ce qui permettrait de dynamiser les débats au sein des conseils qui, chacun le sait, ne sont pas toujours très fournis.

Il est grand temps de marquer un coup d'arrêt à cette entreprise dont la poursuite éloignerait encore un peu plus les Français du jeu démocratique.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, avant tout, je tiens à saluer l'initiative de notre collègue Mireille Jouve et du groupe du RDSE. Elle nous permet aujourd'hui d'avoir de nouveau un débat sur une question majeure pour l'organisation de notre maillage territorial, l'élection des conseillers métropolitains, qui soulève évidemment celle du lien particulier entre communes et métropoles. Mireille Jouve, ancienne maire de Meyrargues, belle commune rurale du Pays d'Aix, connaît bien les problèmes de démocratie que peuvent rencontrer les communes au sein des assemblées métropolitaines. territoire où la création de la métropole Aix-Marseille Provence a été imposée contre l'avis de 113 maires sur 118 et continue d'être rejetée avec force. Considérons la résistance du Pays d'Aix, mais aussi celle du Pays d'Arles, prêt à changer de département pour ne pas être intégré métropole est rejetée avec force tant elle est budgétairement mortifère : une dette de 2 milliards d'euros, une capacité d'investissement quasiment réduite de moitié en deux ans d'existence, une conception en dépit du bon sens sur un territoire comprenant six intercommunalités, le plus étendu de France. Nous avons vécu de l'intérieur l'écrasement de la voix des communes et pu mesurer aussi combien il était dangereux de ne pas tenir compte de leur avis. Si on les avait écoutées, nous n'en serions pas là, avec 2 milliards d'euros de dette, des conventions de gestion pas toujours régulières, notamment sur la clôture des budgets annexes ou sur les exigences d'évaluation préalable, des conventions de gestion sur l'ensemble des compétences communales transférées à la métropole, laquelle, se trouvant dans l'incapacité de gérer ces compétences, a imposé aux communes de le faire pour son compte. Si les communes avaient été entendues, la métropole aurait peut-être été une métropole de projets, et donc une intercommunalité viable, agréable même et prospère. Paraphrasant Benoist Apparu, je dirai que les gouvernements qui se sont succédé ont cédé à la tentation du « grand » et, n'ayant pu supprimer les communes, ont tenté de les vider totalement de leur substance : voirie, parkings, politique de la ville, eau, assainissement, et j'en passe, jusqu'aux lieux de sépulture Il n'en reste pas moins que les communes sont les racines des métropoles. Si leurs exécutifs demeurent les mieux élus de France, c'est bien parce qu'elles sont seules à assurer un lien de proximité réel, un lien démocratique avec les citoyens. Les intercommunalités ont été créées pour aborder à un niveau supracommunal les grands enjeux territoriaux, comme le développement économique, l'environnement, les transports. Aux intercommunalités, c'est-à-dire aux communes réunies, à l'émanation des communes plus exactement, un regard plus large, de long terme, des projets et des moyens supérieurs aux communes, la vie quotidienne, le contact et ... la sanction démocratique directe. Aujourd'hui, l'élargissement autoritaire des compétences intercommunales n'a plus rien à voir avec la logique de subsidiarité qui a présidé à la création des intercommunalités. Ces grands ensembles visent à prendre la place des communes. Mais, sans ancrage suffisant, cela ne fonctionne pas. Le citoyen ne s'y retrouve pas. Le Parlement a déjà voté huit révisions de la loi NOTRe. La semaine prochaine, pour tenir compte, encore une fois, des réalités de terrain, nous devrons revenir sur la compétence eau et assainissement. Les maires et les élus municipaux exercent leurs mandats dans un esprit de proximité, de connaissance profonde des besoins de leurs concitoyens, et ils ont été élus précisément pour cela : pour être au contact, à proximité d'« engueulades », diraient certains.

prise en considération et l'acceptation d'une grande diversité. L'élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains conduirait à un modèle extrêmement politisé, viderait les communes de leur substance et distendrait encore considérablement le lien entre le citoyen et la décision intéressant son quotidien. de l'élection au suffrage universel remonte à la loi de réforme des collectivités de 2010. Les maires avaient riposté avec force : en conséquence, le Sénat avait changé de majorité pour la première fois dans l'histoire de la V République ; souvenons-nous-en.

Au départ, afin d'être mieux identifiées, quelques communautés urbaines se sont constituées en métropole. Aujourd'hui, avec la fusion des régions et malgré de multiples craintes concernant le régime juridique, les capitales de département, de région ou d'ancienne région y viennent de peur de perdre toute visibilité. L'ambition initiale d'identifier quelques métropoles à dimension européenne, voire mondiale, est bien loin. Reste que 72 % de la population vit en dehors des métropoles ; pour une grande part, ces Français sont ceux Les inégalités se sont dangereusement creusées. Nombre d'ambiguïtés demeurent sur le concept de métropole, qui, dans l'imaginaire collectif, renvoie à d'immenses entités, comme Shanghai ou Mexico : super ville-centre, entité nouvelle, voire non encore bien identifiée ? Il est indispensable de clarifier le débat. Qui, demain, sera élu au conseil métropolitain ? Les membres d'une liste portant une étiquette politique peu représentative des nuances et particularités locales ? Les membres d'une liste qui seront uniquement responsables devant leur président et son cabinet ? Ou bien des élus proches des habitants et risquant une double sanction électorale ? Les métropoles ne sont pas des collectivités territoriales ; elles ne sont pas indépendantes, elles dépendent d'autres collectivités, les communes, tant d'ailleurs par leur périmètre que par leurs compétences. que par leurs compétences. Mme la ministre l'a rappelé, aucune collectivité ne doit dépendre d'une autre ; du moins est-ce le sens de l'article 72 de la Constitution. Élire demain les conseillers métropolitains sans fléchage serait changer la nature de la métropole, mais aussi celle de toutes les communes. de loi est indispensable pour lever l'ambiguïté de l'article 54 de la loi MAPTAM, si bien détaillée par notre rapporteur Agnès Canayer, que je remercie de son travail. Plus de quatre ans après la promulgation de la loi MAPTAM, nous ne pouvons demeurer dans l'incertitude sur l'élection des conseillers métropolitains. Une clarification est indispensable, et la présente proposition de loi la permet. Le Sénat a toujours été opposé à ce que les conseillers métropolitains soient élus selon un mode de suffrage universel direct qui ne reposerait plus sur un ancrage communal. En adoptant cette proposition de loi mercredi dernier, la commission des lois de la Haute Assemblée s'est inscrite dans la parfaite continuité de la position qu'elle avait défendue lors des deux lectures du projet de loi MAPTAM.

Le système actuel du fléchage est le meilleur trouvé à ce jour, le seul respectant tant les citoyens dans leur rôle d'habitants des communes que les principes fondateurs de l'intercommunalité. La métropole lyonnaise est souvent présentée comme le modèle à suivre ; ma collègue Michèle Vullien en parlerait sûrement beaucoup mieux que moi. Son cas est très spécifique et ne peut être comparé à d'autres. Ne nous y trompons pas.

Le modèle lyonnais n'est décidément pas comparable aux autres. Le temps pris pour sa construction a été essentiel et lui a permis d'atteindre une certaine sagesse en termes de cohabitation, au sein d'un pôle métropolitain plus vaste, avec une autre ville-centre plus petite, Saint-Étienne.

au conseil métropolitain, et rien ne garantit que chaque commune y soit représentée fût-ce par un seul élu. C'est là une atteinte grave à la représentation démocratique ; c'est exactement ce que nous craignons et rejetons, madame la ministre.

Ayant entendu parler le Premier ministre hier, je voudrais vous inviter à appliquer la même logique mathématique à ce qui nous est proposé pour le Sénat.

MAPTAM, prévoit que le législateur définisse, avant le 1 janvier 2019, un nouveau mode de scrutin pour l'élection des conseillers métropolitains. Depuis plus de quatre ans, le Sénat s'est opposé à une telle réforme, craignant qu'elle ne remette en cause la commune en tant que cellule de base de la démocratie locale. Dans cette logique, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui tend à confirmer l'actuel mode d'élection des conseillers métropolitains et vise ainsi à abroger l'article 54 de la loi MAPTAM. Au même titre que les autres EPCI à fiscalité propre, les métropoles sont nées d'une volonté de coopération de plusieurs collectivités territoriales qui ont souhaité mutualiser certaines compétences et mener des projets d'intérêt métropolitain. Aussi, procéder à des modifications du mode d'élection des conseillers métropolitains reviendrait à remettre en cause les fondements mêmes de l'intercommunalité. Réformer le mode d'élection des conseillers métropolitains présente deux risques majeurs la transformation des métropoles en collectivités territoriales ; d'autre part, la mort des communes, cellules de base de la démocratie locale. Comment imposer une complexité administrative supplémentaire ? Comment imaginer un nouvel empilement institutionnel ?

Les conseils métropolitains doivent donc rester l'émanation directe des conseils municipaux. Je me réjouis que la commission des lois du Sénat ait adopté sans réserve cette proposition de loi. Considérant qu'il est souhaitable de conserver l'ancrage communal des délégués communautaires, pour qu'ils demeurent les représentants des conseils municipaux dans toutes les intercommunalités, des communautés de communes aux métropoles, le groupe Les Indépendants approuve l'abrogation de l'article 54 de la loi MAPTAM et votera en faveur de l'adoption de cette proposition de loi. La parole est

celui des métropoles. Il nous est proposé d'abroger l'article 54 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ce dont il est question ici, c'est bel et bien du sujet des grandes métropoles, au travers de celui de l'élection de ses conseillers. Que reproche-t-on à l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct ? La même chose que l'on reproche aux métropoles elles-mêmes : l'éloignement des réalités locales et la création d'un doublon administratif non représentatif. Avec les métropoles, vous avez encore créé un échelon administratif supplémentaire, qui étouffe littéralement les élus locaux et dilue toujours plus leur pouvoir décisionnel, pour finalement le leur retirer, alors qu'ils sont au contact des réalités, et donc des besoins de leur population. Vous avez aussi créé de nouvelles sources de dépenses, alors même que les collectivités se trouvent asphyxiées par la baisse des dotations de l'État, ce qui oblige les communes à accroître la pression fiscale locale jusqu'à un niveau confiscatoire, comme à Marseille. La décentralisation désordonnée que nous subissons entraîne une situation déjà intenable, avec des collectivités aux ressources réduites, mais aux compétences larges et aux coûts de fonctionnement énormes. Par exemple, la métropole Aix-Marseille Provence, créée dans l'unique but, nous avait-on dit, de développer les transports et de favoriser l'emploi ainsi que l'activité économique, a très vite dérapé, pour se mêler de tout et de n'importe quoi, depuis la voirie jusqu'à l'entretien des piscines. Les coûts et la dette explosent, et c'est la guerre de tranchées qui s'instaure entre les maires, qui perdent inopportunément leurs prérogatives, et un président de la métropole tout aussi puissant qu'éloigné des réalités locales. définitive, ce sont les habitants qui trinquent deux fois : ils paient davantage pour des services de moins en moins ou mal rendus, avec un décideur désormais inaccessible. L'imbroglio entre toutes les strates de l'échelon administratif est une évidence ; nous l'avions annoncé, il saute désormais aux yeux. La solution trouvée par l'exécutif ? Fusionner, d'ici à 2021, cinq métropoles et départements, dont Aix-Marseille Provence avec les Bouches-du-Rhône. Je m'oppose catégoriquement à cette dilution, qui est un non-sens et bafoue encore une fois chacune des communes de Provence. Contrairement à ce qu'affirment certains, il n'y a ni inéluctabilité ni sens de l'histoire, il n'y a que la volonté d'hommes et de femmes attachés, ou pas, à l'identité politique et administrative de leur pays. Je réaffirme que le Front national souhaite que l'organisation territoriale de la France reste fidèle à son histoire, qui repose sur un pouvoir étatique relativement fort, capable de respecter les autonomies et les particularités locales. Nous rejetons cette vision merkelienne, européiste qui vise à l'uniformisation de nos territoires par le biais de la création de métropoles mastodontes faisant table rase de l'État-nation et retirant aux communes leurs libertés, donc leur identité. leur identité. Maintenir une organisation administrative cohérente, garantissant les particularismes, les identités locales et l'unité nationale au travers d'un triptyque puissant et moderne « communes-départements-État » est un enjeu majeur et une alternative crédible, à laquelle sont attachés les élus locaux et les Français. Pour conclure d'une phrase, en matière d'organisation politique, administrative et électorale aussi, il ne saurait y avoir de modernité qu'enracinée dans la tradition

l'objet de la présente proposition de loi est, comme nous en rêvions, clair et simple. Son article unique permettra d'apporter une réponse concrète et pragmatique, dès les élections municipales prochaines de 2020, à la question de l'élection simultanée des conseillers métropolitains.

Sur ce sujet, je suis intimement convaincue que, au-delà du récurrent et légitime débat sur les compétences de nos collectivités, la question des modalités de l'élection des conseillers métropolitains n'est pas accessoire. Bien au contraire,

assume le sien en conscience. Soit nous nous acheminons, ainsi que la loi MAPTAM en dispose, vers la désignation des conseillers métropolitains par le biais d'un scrutin autonome, d'une élection à part entière, déconnectée de l'élection communale, dont il appartient au Gouvernement de définir encore les modalités ; soit nous restons dans le cadre du système actuel de fléchage, qui a démontré, par défaut mais sans défaut, toute sa pertinence. Ce mode de scrutin, contrairement à ce que nous entendons dire parfois, n'est aucunement un déni de démocratie. La forme- un seul bulletin au lieu de deux -ne doit pas nous faire oublier le fond : le système de fléchage est bien un scrutin au suffrage universel direct ; il répond donc aux exigences démocratiques qui nous animent toutes et tous ici. Pour aller plus avant et vous dire le fond de ma pensée, j'estime qu'il est tout simplement inconcevable que les métropoles de droit commun se transforment en collectivités territoriales à statut particulier. Cette conviction, je la tiens de mon expérience de conseillère métropolitaine à Bordeaux. L'intercommunalité doit demeurer une strate de projets, de coopération et d'investissements sur des dossiers structurants à l'échelle métropolitaine ; elle ne peut remplacer le fait communal. À Bordeaux, l'intégration renforcée au sein de la métropole prend la forme d'une mutualisation des services supports, plus ou moins poussée en fonction du choix des communes de conserver, ou pas, certaines compétences. Cela fonctionne très bien ainsi. de dire qu'il est erroné, ou un brin fallacieux, d'affirmer que le système actuel fait disparaître la métropole du débat électoral. Au contraire, le fait métropolitain s'impose à nous : c'est une évidence dans les vingt-deux territoires concernés. Qui oserait prétendre le contraire ? Cessons de faire croire que le débat qui a lieu lors des campagnes municipales serait uniquement centré sur les « bouts de trottoir » de nos administrés. Ce n'est pas vrai, et nos concitoyens le savent : quand un campus d'excellence s'installe, quand de grandes entreprises s'implantent, quand il s'agit de doter une métropole d'un pont, d'un stade ou d'une « arena », nous savons tous que nous parlons de l'intercommunalité. La métropole est donc l'échelon du projet, de l'infrastructure, mais aussi cet acteur qui s'ouvre vers l'extérieur, qui engage le dialogue avec les villes d'équilibre, qui parle aux agglomérations, qui contractualise avec les territoires de son écosystème le plus en difficulté. Il y a cependant un préalable de gouvernance : la métropole doit mettre les élus de toutes les communes qui la composent autour de la table, et plus précisément leurs maires. Nous sommes là au coeur du fondement du pacte intercommunal. C'est un prérequis indispensable à une gouvernance qui privilégie le dialogue : dialogue entre les élus, mais aussi dialogue entre les services, rendu possible parce que le maire de la commune siège à la métropole et qu'il y est considéré, écouté et entendu. Nous refusons la généralisation automatique d'un système « à la lyonnaise », où certains maires inaugureraient les chrysanthèmes dans leur commune, mais ne seraient pas représentés au sein de la métropole. La représentation des communes n'est pas négociable Mes chers collègues, vous l'aurez compris, cette proposition de loi vise à défendre la place de la commune, fruit de la légitimité et de la longévité de l'histoire républicaine de notre pays. Quant à l'intercommunalité, laissons-lui la place qui est la sienne, c'est-à-dire le prolongement direct des enjeux municipaux et la résultante d'un pacte politique pour le territoire, autour d'un projet partagé. métropoles ne rentrent pas dans des cases. Elles ont leurs spécificités, qu'elles soient de taille européenne ou de taille plus modeste, qu'elles soient administrées dans une logique de cogestion, comme à Bordeaux, ou selon un autre mode de gouvernance.

L'idée du scrutin supra-communal est donc contradictoire. Elle ne pourrait être satisfaite qu'à travers un système qui transformerait l'intercommunalité en collectivité, avec une série de conséquences fâcheuses,

ministère de l'intérieur ... - et une possibilité d'évolution dans la relation administrative entre les communes et l'intercommunalité. Si l'on crée une intercommunalité qui devient une collectivité pour elle-même, cette fluidité n'existe plus.

pays. Premièrement, il n'a pas l'intention de proposer une nouvelle grande réorganisation territoriale, préférant amortir celles qui ont eu lieu.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, si notre collègue Jean-Pierre Sueur voit dans ce texte une précaution inutile,

avons la conviction profonde que la commune est la cellule de base de la démocratie française et la porte d'entrée vers l'intercommunalité, laquelle doit rester un espace de projets et de mutualisation. Oui, nous réaffirmons notre attachement à la commune. Au moment où nos concitoyens nous demandent

de Strasbourg. Les communes doivent être défendues. En même temps, elles se défendent mieux lorsqu'elles sont dans des intercommunalités renforcées,

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui présente l'avantage de ménager une pause dans les réformes de l'organisation territoriale, pause qui est souhaitée par les élus locaux- et c'est le rôle c'est le rôle du Sénat d'être à l'écoute de ces derniers. Selon le droit en vigueur, les conseillers métropolitains sont désignés à l'occasion des élections municipales, soit par le système du fléchage dans les communes de 1 000 habitants et plus, soit selon l'ordre du tableau du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Ce mode de désignation permet de respecter les principes fondamentaux qui régissent la composition des conseils communautaires, comme la participation de toutes les communes membres ou la représentation des citoyens sur des bases essentiellement démographiques. Par ailleurs, grâce au système de fléchage, plus de 95 % des conseillers métropolitains sont d'ores et déjà élus au suffrage universel direct. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ou loi MAPTAM, est source d'ambiguïté. En effet, son article 54 a créé l'incertitude en demandant au législateur de définir, avant le 1 janvier 2019, les modalités de l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. Le rapport remis par le Gouvernement trois ans après l'adoption de cette loi dégage trois pistes de réflexion. Le premier scénario prévoit la coexistence de deux collèges distincts au sein d'un même conseil métropolitain. Dans le deuxième scénario du Gouvernement, les conseillers métropolitains resteraient élus dans des circonscriptions communales, mais les élections municipales et métropolitaines seraient dissociées. Enfin, le troisième scénario apparaît proche du scrutin existant pour les conseils régionaux : le conseil métropolitain serait élu à la représentation proportionnelle avec une prime majoritaire, dans une circonscription unique, mais avec des sections électorales communales. Que d'ambiguïté ! Madame la ministre, mes chers collègues, au système actuel d'élection des conseillers métropolitains, je préférais pour ma part le précédent, qui laissait la souplesse aux conseils municipaux de désigner de nouveaux représentants au sein des conseils communautaires en cours de mandat. Par exemple, un maire nouvellement élu est dans l'impossibilité de siéger au conseil communautaire dans la mesure où il ne figurait pas dans le fléchage.

Je remarque tout d'abord que les métropoles sont de nature très diverse. Comment comparer les onze métropoles de droit commun correspondant à des EPCI à fiscalité propre de 400 000 habitants dans une aire urbaine de 650 000 habitants-

Sophie Joissains nous a décrit le fonctionnement, voire les dysfonctionnements, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. En tant qu'élue de la métropole du Grand Paris au titre de mon mandat à Boulogne-Billancourt et dans l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, je vous parlerai de la métropole du Grand Paris. du Grand Paris. Je le rappelle, cette « métropole » a été bâtie contre l'avis des maires et des élus locaux, qui se sont prononcés à deux reprises contre les textes MAPTAM et NOTRe au sein de la mission de préfiguration du Grand Paris à plus de 75 % en octobre 2013 et à 94 % en octobre 2014. J'ai bien entendu les propos d'Alain Richard, qui, reprenant les intentions du Président de la République, a évoqué des évolutions volontaires pour six ou sept grandes métropoles. Aujourd'hui, évoquer la métropole du Grand Paris, c'est faire une sorte de « voyage en Absurdie », sur le plan institutionnel comme sur le plan financier. Elle n'exerce pas de véritables compétences opérationnelles, mais suscite 3,4 milliards d'euros de flux financiers, pour un budget primitif pour 2018 de 29,3 millions d'euros après retraitement des flux entre la métropole et les communes, soit moins de 4,3 euros par habitant pour fonctionner. L'épargne brute de cet ensemble de plus de 7 millions d'habitants est de seulement 5 millions d'euros.

Faute de projet, la métropole du Grand Paris a investi seulement 16 millions d'euros en 2017. Les territoires, qui ont dû transférer une partie de leur fiscalité économique à la métropole, auraient su mobiliser utilement la croissance de la CVAE du territoire francilien au bénéfice de l'économie nationale. Privés de leurs moyens financiers, ils ont dû geler des investissements programmés et proches des citoyens. En l'état, une élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains du Grand Paris, détachée des communes, serait une catastrophe, sauf à vouloir en faire une sorte de « super-département » intercalé entre les blocs communaux et la région. Une nouvelle couche supplémentaire à un millefeuille déjà bien indigeste Madame la ministre, alors sénatrice du Loir-et-Cher, vous aviez justement fait remarquer, dans le cadre de l'examen d'un amendement déposé lors de la seconde lecture de la loi MAPTAM, qu'élire les conseillers métropolitains au suffrage universel direct reviendrait, de fait, à créer une nouvelle collectivité territoriale. Par ailleurs, quelle cohérence y aurait-il à définir aujourd'hui les modalités d'élection d'élus dont on ne connaît toujours pas les attributions dans les prochaines années ? Le Président de la République, qui a déjà repoussé à plusieurs reprises ses annonces sur la réforme du Grand Paris, prendra-t-il conscience que, tant qu'il ne se sera pas prononcé, l'incertitude et le flou institutionnel continueront de régner, rendant impossible toute action et toute gestion saine de nos collectivités ? Le mode d'élection actuel des conseillers métropolitains par fléchage permet de maintenir un lien de proximité entre les citoyens, les élus locaux et leurs représentants au sein de l'échelon métropolitain.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur,

de moderniser les territoires et d'assurer leur développement économique. Ce nouveau concept marque des points, mais il rencontre aussi des problèmes dans son application au quotidien.

qui reste l'interlocuteur direct des administrés. Or l'article 54 de la loi MAPTAM pourrait appauvrir les relations territoriales et amplifier les concurrences institutionnelles. Dans l'intérêt des habitants, il faut préserver l'équilibre structurel des collaborations horizontales qui existent actuellement entre les communes membres et les métropoles. Conseiller métropolitain lyonnais, je suis attaché à une action publique plus efficace, plus rapide et plus cohérente pour la vie quotidienne de nos territoires.

n'aurait plus de prise sur la décision et ne pourrait même pas donner un avis sur des travaux réalisés sur son territoire. À l'occasion de ce débat, avec mes trois collègues sénateurs Les Républicains et apparentés du Rhône, François-Noël Buffet, Élisabeth Lamure et Catherine Di Folco,

Nous voulions engager le débat sur les relations entre la métropole de Lyon, les maires et les conseils municipaux dans la nouvelle donne de 2020.

Ces délégations doivent être fixées dans le cadre du pacte de cohérence métropolitain qui est rédigé à chaque début de mandat,

ainsi ! Très bien ! La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette initiative parlementaire de nos collègues du groupe du RDSE ouvre le débat sur l'élection des conseillers métropolitains. Le 1 janvier 2015, l'agglomération de Montpellier une métropole. Cette expérience m'autorise aujourd'hui à porter ici, au Sénat, le témoignage d'un EPCI qui fonctionnait parfaitement jusqu'à sa transformation. Pour ma part, j'avais appelé de mes voeux cette évolution, dès lors que le gouvernement précédent nous garantissait une transformation en métropole librement consentie par les communes, et non effectuée un simple décret, une dotation financière spécifique pour les nouvelles métropoles et un mode de représentation des communes qui restait directement lié au résultat de l'élection municipale dans chaque commune.

Aussi, chacun comprendra que je souscrive à l'objet de cet article unique. J'avais déposé un amendement identique lors de l'examen, en novembre dernier, de la proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections. Toutefois, cet amendement avait alors été déclaré irrecevable. Dans son rapport de janvier 2017, le précédent gouvernement constatait l'absence de consensus politique en la matière. Il semblait néanmoins privilégier l'hypothèse d'une assemblée élue dans le cadre d'une circonscription unique dotée de sections électorales. Ce mode de scrutin Ce mode de scrutin pose un problème majeur quant au respect de la démocratie. À titre d'exemple, dans les sections communales ne comportant qu'un seul siège, un candidat issu d'une liste arrivée en tête à l'échelle de la métropole pourrait être élu dans sa section communale, en application de la prime majoritaire, alors que, dans cette même commune, la liste arrivée en tête n'aurait pas de représentant.

cher collègue. ... pourrait ne plus être le maire, mais un conseiller de l'opposition, voire une personne extérieure au conseil municipal. Or la logique de l'intercommunalité veut que le conseiller métropolitain soit un représentant de sa commune,

ou loi NOTRe, a tenté de les faire disparaître ; les baisses inouïes de dotations décidées pendant le précédent quinquennat les ont rudement malmenés ; enfin, la perte programmée de toute autonomie financière à la suite de la disparition de la taxe d'habitation, inexorablement suivie de la part départementale

Si les métropoles se saisissaient des compétences départementales dans leurs territoires, qu'adviendrait-il du reste ? L'espace départemental non métropolitain, cet arrière-pays vital pour les habitants des métropoles, serait abandonné à lui-même, sans ressources en proportion de ses besoins. ne serait plus que l'ultra-périphérie de la France périphérique ! Il suffit d'écouter le président du conseil départemental du Rhône pour s'en convaincre. L'élection des conseillers métropolitains

sur l'article unique. Mes chers collègues, la commune est la cellule de base de la République. Elle est le premier lieu d'expression de la démocratie, de recueil de la demande sociale, de décision et d'exécution pour apporter des solutions aux problèmes concrets des habitants.

des syndicats de communes aux EPCI d'aujourd'hui, de la communauté de communes à la métropole. Aujourd'hui, si les intercommunalités fonctionnent bien, c'est parce qu'elles procèdent des communes. Cette symbiose avec les communes membres est la condition du bon il faut que les communes soient entendues, que les maires portent la voix de leur commune dans l'intercommunalité et, souvent, que l'exécutif de cette dernière cultive une forme de collégialité avec les maires.

repose sur une condition fondamentale : l'élection des conseillers métropolitains dans la circonscription communale. Le mode de scrutin direct est déjà assuré par le fléchage, par ces bulletins de vote « deux en un » que nous avions imaginés pour nous conformer au principe constitutionnel tout en restant dans la circonscription communale et en maintenant le lien entre l'exécutif municipal et la représentation de la commune dans l'EPCI.

et le bon fonctionnement de nos métropoles. Il est temps de stabiliser la situation des communes au sein des métropoles, afin que les métropoles et les communes puissent travailler sereinement

y être représentées et pouvoir s'y exprimer. Néanmoins, la méthode d'élection actuelle des conseillers métropolitains, pour la très grande majorité par fléchage, n'est pas satisfaisante : qui pourrait dire le contraire ? Aussi, nous devons tirer parti de ce débat. Le ne va pas dans le sens de l'histoire, bien au contraire.

ce qui garantirait la représentation de chaque commune au sein du conseil métropolitain. Le tiers restant serait élu au suffrage universel direct dans le cadre d'une circonscription métropolitaine unique, ce qui permettrait aux citoyens de s'exprimer aux projets métropolitains et d'en débattre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce scrutin serait régi par les mêmes règles que les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus. Je précise que nous avons modélisé

La loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a, par son article 78, repoussé au 1 janvier 2019 l'adoption d'une loi définissant le cadre applicable à l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct.

Ce faisant, le prochain renouvellement des conseils municipaux s'organiserait selon le mode d'élection actuel. Au regard des crispations suscitées par la pérennisation d'un scrutin distinct de celui qui désigne les élus municipaux, les dispositions de cet amendement s'inscrivent dans une démarche constructive.

! Est-ce que renforcer encore, par le mode de scrutin, le poids des communs centres et des plus grosses communes permettra de développer la démocratie ? Pas du tout !

sur le texte dont vous êtes l'auteur, chère Mireille Jouve, est d'apporter une clarification nécessaire sur les intentions du Gouvernement. Nous sommes nombreux dans l'hémicycle à considérer que cette clarification était utile et à en remercier Mme Gourault, qui s'est exprimée

des conseillers départementaux a rendu incompatible le mandat de conseiller communautaire avec un emploi salarié au sein d'une des communes membres. Or le mandat de conseiller municipal au sein d'une des communes membres n'est, lui, pas incompatible avec un emploi salarié au sein de l'intercommunalité.

En repli, l'amendement n° 2 tend à prévoir un mécanisme permettant à l'élu de retrouver son mandat de conseiller communautaire dès que cesse l'incompatibilité.

Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus pour la première fois par fléchage sur les listes de candidats au conseil municipal dans les communes de plus de 1 000 habitants. Les principaux objectifs de la réforme de 2013 étaient de renforcer la parité, d'améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités et de rendre leur fonctionnement plus lisible pour les citoyens. Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas. En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale. Les aléas de la vie municipale font qu'un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale en cours du mandat. La commune peut alors être représentée par un ex-élu de sa majorité, celui-ci se pouvant même se voir confier des responsabilités dans l'exécutif intercommunal. Afin de maintenir une stabilité municipale, cet amendement d'appel

de la majorité municipale s'étant fâché avec le maire, le président de la métropole de Montpellier a destitué le maire de ses fonctions de vice-président et a mis son opposant à sa place. La démocratie est bafouée ! L'amendement n° 6, Jean-Pierre Grand. Pour les communes de plus de 1 000 habitants, la loi du 17 mai 2013 a fixé de nombreuses règles pour la présentation de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire. La complexité de ces règles les candidats de toute souplesse dans l'élaboration de leur liste. Aussi, il est proposé de supprimer l'obligation de faire figurer les candidats dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil

Jean-Pierre Grand. Mes chers collègues, si la Haute Assemblée décide de ne pas revenir sur le système de fléchage pour l'élection des conseillers communautaires, je vous propose d'instaurer une clause de rendez-vous permettant aux communes disposant d'un nombre de conseillers inférieur dixième de l'effectif total du conseil communautaire de procéder à la désignation de nouveaux conseillers au cours du mandat. Cette nouvelle désignation devra bien sûr respecter la répartition du nombre de sièges et la répartition selon le sexe des candidats établies entre les listes lors de la

Or cette contrainte n'a pas de réelle justification. En effet, il n'existe aucun lien entre la composition d'un exécutif municipal et les compétences de l'intercommunalité. Durant mon mandat de maire de presque trente-cinq ans, mes trois premiers adjoints successifs étaient délégués à l'action sociale. Selon quel principe un maire devrait-il définir l'ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l'intercommunalité ? Au contraire, pour une plus grande souplesse, il conviendrait de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation. Madame la ministre, je ne résiste pas au plaisir de rappeler que

dans les communes qui disposent d'un nombre de conseillers communautaires inférieur au dixième de l'effectif du conseil municipal. Un tel dispositif me semble complexe à mettre en oeuvre.

Certes, mais en connaissez-vous un autre qui permette de satisfaire l'ensemble des critères et des contraintes rappelés tout à l'heure par Mme la ministre ? Non !

et c'est pour cela que, bien que ne doutant aucunement de l'issue d'un vote à main levée, j'ai demandé un vote par scrutin public. Chacun prendra ses responsabilités

de la métropole de Lyon, en charge précisément de la mise en place de cette nouvelle entité. Je puis témoigner du bien-fondé de la construction métropolitaine, qui a été le mariage de l'humain et l'urbain et qui a supprimé une couche du millefeuille administratif. En revanche, je puis également témoigner du refus par les élus métropolitains du mode de scrutin prévu en 2020, qui va priver certaines communes d'une représentation au conseil de la métropole de Lyon,

cet échelon qui est rassurant pour l'habitant qui a tout à perdre s'il est livré au bon vouloir de la technostructure. On voit d'ailleurs poindre à l'horizon la disparition pure et simple de la commune-certains collègues ne s'y sont pas trompés. Nous alertons depuis plus de quatre ans sur les conséquences néfastes pour les communes et leurs habitants. La métropole de Lyon devait servir de modèle aux autres métropoles françaises. Or que se passe-t-il ?

cette vision. Aussi voterai-je la proposition de loi, en lançant un cri d'alarme pour l'avenir : nous risquons bien de voir disparaître l'échelon communal au profit d'une technostructure très éloignée des besoins réels du citoyen ! Il est clair que le mode électoral de la métropole de Lyon devra également être revu,

était besoin, que l'avenir des métropoles suscite débats et intérêt. Lucides, nous nourrissons un espoir mesuré de voir ce texte repris et adopté par les députés. Néanmoins, nous pouvons nous féliciter de la suppression de l'article 54 de la loi MAPTAM. Elle nous permet, comme Mme la rapporteur l'a souligné, de sortir de l'ambiguïté et de l'impasse.

Je serais tentée de lui répondre que c'est l'article 54 qui a fait la preuve de son inutilité ! De fait, celui-ci prévoit la remise d'un rapport rendu avec plus d'un an et demi de retard et demande au Gouvernement de légiférer sans que cette disposition ait de valeur normative.

sans les communes, ni contre les communes. Or les échos des négociations et tractations en cours dans les cinq métropoles de taille européenne sont de nature à inquiéter, car les communes sont mises hors-jeu. Nous pensons que la force de l'intercommunalité est de reposer, comme l'indique le sigle « EPCI », sur la coopération. Nous sommes nombreux à estimer aussi que la situation n'est pas mûre pour une évolution du mode de scrutin et que nos métropoles ont besoin de stabilité pour grandir et assumer pleinement leurs compétences. Mme la ministre nous a annoncé que nous serons amenés à débattre d'un projet de loi prévoyant la transformation de cinq à huit métropoles en collectivités à statut particulier, en rupture avec le modèle de la coopération intercommunale. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Personne ne

Le scrutin est ouvert.

mes chers collègues,

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. L'orateur du groupe qui a demandé ce débat disposera d'un temps de parole de dix minutes, y compris la réplique, puis le Gouvernement répondra pour une durée équivalente.

Les problématiques touchant à la médecine, à la répartition territoriale des praticiens et à l'avenir de notre système de santé prennent une place croissante dans nos travaux et dans la société. La santé est devenue l'une des toutes premières préoccupations des Français. Le groupe du RDSE, toujours sensible aux questions de santé publique et de maillage territorial, a souhaité mettre à l'ordre du jour ce débat, qui nous permet de prendre une part active à la concertation sur la réforme des études médicales lancée en mars dernier par le Gouvernement. La formation des médecins et les ressources humaines sont un pilier essentiel de la transformation de notre système de santé. Celle-ci intervient dans un contexte de grandes difficultés d'accès aux soins et d'une certaine désaffection des praticiens, associés à un profond malaise des étudiants. Confrontés à un double carcan- le en fin de première année et les épreuves classantes nationales, ou ECN, en fin de deuxième cycle -les étudiants en santé sont soumis à des conditions de vie dégradées, comme l'a souligné dans son rapport le professeur Diot, président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé. Une vaste enquête sur la santé mentale des jeunes médecins, menée l'année dernière par l'Association nationale des étudiants en médecine de France, le confirme : plus des deux tiers des carabins présentent des symptômes anxieux, un tiers des symptômes dépressifs et un quart des idées suicidaires, avec des passages à l'acte malheureusement trop fréquents. La moitié des étudiants en médecine ont déjà songé à arrêter leur cursus. Ces résultats sont accablants ! Quelques pistes peuvent expliquer ce malaise : un cursus excessivement sélectif ; une charge de travail très lourde, avec une réglementation européenne sur les quarante-huit heures hebdomadaires et le repos de sécurité qui n'est, hélas, pas toujours respectée ; la confrontation à la maladie et à la mort ; une trop grande responsabilisation d'étudiants pas toujours bien préparés ; des conduites de management inappropriées, avec encore des situations de harcèlement, de pression, voire de sexisme. Ce malaise doit être entendu. Si de telles conditions de vie et d'apprentissage pouvaient jusqu'ici être tolérées, aujourd'hui, la situation n'est plus acceptable. Nous saluons donc les engagements pris avant-hier

Le, défini comme un outil de régulation, montreses limites et doit, à de nombreux titres, être repensé. Il est d'abord inefficace en ce qui concerne la répartition des médecins sur les territoires. Ensuite, son inertie est grande. il est contourné par l'arrivée de médecins étrangers ou de médecins français ayant réalisé leurs études à l'étranger. Enfin, il entraîne un taux d'échec sans alternative qui n'est pas acceptable. Après deux tentatives, en effet, nombre d'étudiants se retrouvent sans rien. On ne peut se satisfaire d'un tel gâchis.

favoriser les alternatives dans un parcours LMD apparaissent comme des solutions intéressantes pour diversifier les profils et éviter le gâchis de la PACES. À la fin du deuxième cycle, l'orientation des futurs médecins est conditionnée par le classement aux ECN. Leur choix, parfois contraint par ce résultat, les engage dans l'exercice d'une spécialité tout au long de leur carrière, sans réelles possibilités de réorientation.

Après le fiasco des ECN en 2017, le président de la Conférence des doyens de médecine a préconisé leur suppression sous leur forme actuelle, pour privilégier le contrôle continu avec une modulation régionale adaptée aux besoins des territoires et aux capacités de formation des universités. concerne le contenu pédagogique, une plus grande professionnalisation dès le deuxième cycle, une plus grande porosité entre les différentes spécialités et des passerelles au cours des études et de la carrière sont également à envisager. la réforme des études de santé offre une belle occasion de former les étudiants aux nouvelles pratiques et répondre aux enjeux de la médecine d'aujourd'hui. Cela suppose de mettre l'accent, le plus tôt possible, sur le travail en équipe. l'une des premières solutions est l'« universitarisation » des formations de santé : ensemble, sur les bancs de l'université, les étudiants pourront apprendre à coopérer, notamment dans le cadre de temps de formation communs. Un autre souhait des professionnels de santé est d'inciter les étudiants à effectuer plus de stages d'externat, dès le deuxième cycle, en dehors des CHU, dans les hôpitaux périphériques, en maison et pôle de santé, dans le privé comme dans le public et pour toutes les spécialités. la formation encore trop « hospitalo-centrée » et « CHU-centrée » biaise les orientations professionnelles des jeunes médecins. Ces stages leur permettront de mieux appréhender la pratique de la médecine ambulatoire et de mieux connaître les professionnels de santé qui interagissent autour du patient. À n'en pas douter, ils favoriseront les installations futures sur les territoires. Nous saluons les mesures prises en ce sens dans la réforme du troisième cycle, mais un effort considérable reste à faire sur nos territoires en tension en direction des maîtres de stage universitaires, sans quoi les bonnes intentions ne pourront pas se concrétiser. Le médecin de demain, c'est aussi celui qui sait tirer profit des avancées technologiques. Les formations doivent intégrer de nouveaux outils tels que l'« e-santé » et les apports de l'intelligence artificielle. Il est indispensable que la France, qui se veut à la pointe dans ce domaine, laisse toute sa place à l'innovation, que celle-ci soit technologique ou organisationnelle, dès les études médicales. il paraît indispensable de mieux former les jeunes à la gestion administrative de leur futur travail, car leur impréparation peut être un frein à l'installation. Pour finir, j'aborderai la question des origines sociales et territoriales des étudiants en médecine. D'après une étude, quatre étudiants sur dix de la PACES 2013-2014 venaient de milieux favorisés, ce qui place les études de santé parmi les formations les plus clivées socialement. La même étude a montré qu'un enfant de cadre avait 2,5 fois plus de chances qu'un enfant d'ouvrier d'intégrer une deuxième année. Ce manque de diversité, difficilement acceptable pour les élus de la République, a, de plus, des conséquences majeures sur l'installation des jeunes praticiens une fois leur diplôme obtenu. Dans ce domaine, des expérimentations intéressantes se déroulent sur notre territoire. Ainsi, dans le Centre-Val de Loire, le parcours « Ambition PACES » vise à susciter des vocations chez des élèves de quatorze lycées ruraux : professeurs et étudiants en médecine proposent un « tutorat santé », en faisant le pari qu'une partie qu'une partie de ces futurs médecins s'installeront sur leur territoire d'origine. Le bénéfice est double, puisque ce dispositif renforce l'égalité des chances. L'inégalité d'accès aux soins nous interpelle tous, et la réforme des études médicales doit répondre à cet enjeu. Devant l'urgence de la situation, certains pensent que la coercition pourrait être une solution. À titre personnel, je ne partage pas cet avis. Des erreurs d'aménagement du territoire ont été commises : trente années d'un mal régulé et, surtout, un manque d'anticipation de la transformation de notre société ont abouti à la situation que nous connaissons. Les incitations financières, nous l'avons vu, ont également leurs limites. Les nouvelles générations de médecins cherchent avant tout un projet pluriprofessionnel, compatible avec un projet familial, sur un territoire où ils se sentent bien. Les collectivités territoriales ont à cet égard tout leur rôle à jouer dans l'accompagnement de cette réforme, par exemple par le soutien aux maisons de santé pluriprofessionnelles ou aux maisons des internes, projets expérimentaux engagés sur mon territoire.

Enfin, il faudrait généraliser, sur les territoires en difficulté, les postes de médecins adjoints, occupés par des étudiants en cours de troisième cycle. Madame la ministre, mes chers collègues, le sujet est vaste, mais les ressources ne manquent pas. Pour améliorer la prise en charge de nos concitoyens, la qualité de vie de nos praticiens et le système de santé publique dans sa globalité, une refonte des formations en santé, avec une attention particulière portée aux étudiants, nous paraît inévitable. Des expérimentations locales existent, qui sont source d'espoir. Nous attendons notamment de la grande concertation qui débute

dès notre arrivée aux responsabilités, l'été dernier. Elles devront prendre en compte les enjeux d'orientation et de réussite des étudiants, de qualité de la formation, de prospective des métiers de demain et de régulation démographique des professions de santé, dans la perspective de répondre aux besoins de la population. Nous avons souhaité, dès le début du quinquennat, revoir l'approche de l'accès aux soins sur le territoire, en agissant dès la formation des futurs professionnels de santé. C'est pourquoi le Premier ministre et moi-même avons présenté, dès le mois d'octobre dernier, un vaste plan d'action pour l'accès territorial aux soins, qui constitue l'un des axes de la stratégie nationale de santé. plan vise à permettre à chaque citoyen d'avoir accès à une médecine de qualité, quel que soit l'endroit où il vit. Il comporte un panel de solutions adaptables à chaque contexte local, car la réponse aux difficultés démographiques n'est pas unique. porteur d'un changement de paradigme, car l'installation de professionnels de santé ne constitue pas la seule action à envisager : tous les leviers de nature à projeter du temps médical dans les territoires et les zones en tension sont à mobiliser.

est encore marquée par un très fort « hospitalo-centrisme ». Il convient donc d'augmenter le nombre de maîtres de stage et d'améliorer l'organisation des stages. C'est pourquoi nous avons proposé que la rémunération des maîtres de stage soit bonifiée pour les médecins installés en zone sous-dense 300 euros supplémentaires par mois, en plus des honoraires de base de 600 euros. Des réflexions sont également en cours afin de faciliter les procédures d'agrément des maîtres de stage. Par ailleurs, il est essentiel que les étudiants puissent être formés dans des lieux d'exercice plus proches de leur exercice futur. Pour permettre ce déploiement des étudiants dans les territoires, une prime à destination des internes qui choisissent d'effectuer un stage ambulatoire en zone sous-dense va être créée : d'un montant de 200 euros par mois, elle sera destinée aux internes qui ne se verront pas proposer par une collectivité territoriale une solution d'hébergement ou une aide à l'hébergement de proximité. Je souhaite que puisse être étendue aux zones sous-denses la possibilité de donner le statut de médecin adjoint aux étudiants en médecine remplissant les conditions pour obtenir une licence de remplacement. Cette possibilité, que vous avez mentionnée, madame Guillotin, était jusqu'à présent limitée aux cas d'afflux exceptionnels de population. Elle permettra de renforcer le temps médical disponible dans des zones identifiées comme prioritaires, en même temps qu'elle permettra à de futurs médecins de s'aguerrir à un certain type d'exercices et, pour certains, de poser les bases de leur projet professionnel. que la répartition des professionnels sur le territoire, si elle est un enjeu essentiel, ne doit pas être le seul objectif d'une réforme des formations de santé.

au contournement européen, avec la reconnaissance automatique des diplômes des médecins formés au sein de l'Union européenne. Je pense aussi au gâchis humain suscité par le concours de la première année, qu'à la hiérarchisation et la stigmatisation des professionnels de santé aux dépens du développement d'un esprit de coopération et de collaboration. Une réflexion a été lancée dans le cadre de la transformation du système de santé ; elle sera sans tabou. De premières propositions nous seront remises, à Frédérique Vidal et à moi-même, à la fin du mois de mai prochain. La première année commune des études de santé doit aussi être réformée, en lien avec les expérimentations d'alternatives lancées par la loi de juillet 2013. La mise en place de la PACES, en 2009, répondait à la volonté de faire face aux conséquences des échecs des candidats. Aujourd'hui, le constat est fait que la PACES n'atteint pas cet objectif et qu'il est nécessaire de la faire évoluer. Les expérimentations lancées visent à répondre à deux objectifs prioritaires : diversifier les profils des étudiants accédant à ces filières ; permettre aux étudiants non admis dans ces filières de poursuivre leurs études en capitalisant sur leur année ou leurs deux années de PACES, sans sans avoir nécessairement à se réinscrire en première année dans un autre cursus. Les expérimentations de ce type ont besoin de temps pour que l'on puisse en mesurer pleinement les effets et les évaluer de façon complète, avant de décider ou non leur généralisation.

Toutes ces expérimentations feront l'objet d'une évaluation que le Gouvernement présentera au Parlement, et nous en tirerons les conséquences qui s'imposent. Le modèle de réforme du deuxième cycle des études de santé doit être repensé, pour permettre de sortir des écueils créés par les épreuves classantes nationales. Ces épreuves de fin de sixième année ont en effet montré leurs limites, et il nous faut repenser le second cycle des études de médecine dans son ensemble. Nous avons confié au professeur Jean-Luc Dubois Randé et au docteur Quentin Hennion-Imbault une mission pour analyser les options possibles. Ils ont remis leurs propositions à fin du mois de décembre dernier. Elles nécessitent un approfondissement, tant certaines sont restructurantes. La proposition la plus marquante est la fin des ECN, qui sont insuffisamment discriminantes, favorisent l'apprentissage théorique et, surtout, ne permettent pas l'appariement entre la compétence et la spécialité. J'ai demandé que ces propositions, qui s'inscrivent dans la continuité de la réforme du troisième cycle des études de médecine, fassent l'objet d'une grande concertation, lancée en mars dernier et qui doit se conclure à l'automne. Ces travaux devront permettre aux formations de donner les clefs nécessaires aux professionnels pour s'adapter aux enjeux du système de santé de demain. demain. La réforme du troisième cycle des études médicales, soit l'internat, avait été rendue nécessaire par l'évolution de la médecine, l'émergence de nouveaux savoirs et pratiques et l'évolution des spécialités. Cette réforme, réalisée en 2016, est porteuse d'avancées pédagogiques concernant l'évolution des pratiques médicales et des outils pédagogiques mobilisables. Elle est toujours en phase de déploiement et fait l'objet d'un suivi approfondi des services du ministère.

En 2017, les études menées par les syndicats et les fédérations d'étudiants en médecine et en soins infirmiers ont mis l'accent sur des situations de maltraitance. Aujourd'hui, il apparaît que, en moyenne, deux tiers des étudiants souffrent d'anxiété ; vous avez donné le chiffre, madame la sénatrice, et je n'y reviens pas. avons donc confié, en juillet dernier, une mission au docteur Donata Marra sur la qualité de vie au travail des étudiants en santé, dans un contexte où les enquêtes et témoignages se multipliaient. Ce rapport met en avant le caractère multifactoriel et complexe de ce mal-être,

d'abord, nous prendrons des mesures immédiates de soutien et d'intervention, en réaffirmant le refus des pratiques inacceptables et en saisissant au besoin les instances disciplinaires. Nous créerons aussi dans toutes les facultés une structure d'accompagnement et nous améliorerons les conditions de travail dans le cadre des stages, par la généralisation des conventions d'accueil des étudiants santé. Nous poursuivrons également la transformation globale des études de santé, en particulier en repensant les cursus pour les centrer sur les compétences à acquérir et sortir d'une logique de compétition. Enfin, nous assurerons des passerelles de sortie avec validation des acquis pour tous les étudiants en santé. Ces chantiers, déjà engagés, doivent maintenant s'articuler les uns avec les autres pour former une évolution cohérente de la formation des médecins de demain, dans une logique plus vaste et de plus longue haleine : celle de la transformation du système de santé. Alors que ce système est en pleine mutation, nous devons nous

Nous devons leur offrir les conditions d'étude qu'ils méritent. Ensemble, nous pouvons agir afin d'adapter les formations et d'anticiper les besoins de demain ! Mes chers

Mais si la compétence des médecins n'est pas en cause, une autre partie du contrat n'est pas remplie aujourd'hui : tous nos concitoyens ne bénéficient pas d'un égal accès aux soins. La situation devient même intenable dans certains territoires qui sont aujourd'hui au bord de la rupture par manque de médecins. Autre problème, le cumul des difficultés dans ces territoires. Près de 20 % des personnes qui vivent dans une commune sous-dotée en médecins généralistes sont éloignées de plus de trente minutes d'un service des urgences. Et la situation est encore plus alarmante s'agissant de l'accès aux médecins spécialistes ! Madame la ministre, ne faudrait-il pas mieux prendre en compte cette réalité lors de la formation des futurs médecins ? Ne faudrait-il pas mieux les informer et les sensibiliser à ces enjeux, favoriser les stages dans les zones sous-dotées, les inciter à s'y installer ou, pourquoi pas, leur proposer une forme de service civique dans ces zones sous-dotées à l'issue de leurs études ? Ne serait-il pas envisageable également de mieux intégrer dans les enseignements l'exercice coordonné entre les différents professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des patients, notamment dans les zones rurales au travers des maisons de santé ? Enfin, je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous redire que, face au décrochage de certains territoires, tant dans l'offre de médecine libérale que dans celle des établissements de santé, il est urgent de prendre des mesures énergiques, de très court terme,

des maîtres de stage dans les zones sous-denses et allons accélérer leur formation. Il existe aussi une prime à destination des internes qui choisissent d'effectuer des stages ambulatoires en zone sous-dense. Nous avons annoncé la création de 300 postes d'assistants partagés ambulatoires

Madame la ministre, mes chers collègues, malgré les initiatives de tous les gouvernements successifs, malgré les aides à l'installation en vigueur, le problème perdure : 2,5 millions de Français vivent encore dans un désert médical en 2018. La formation des étudiants en médecine, leur répartition géographique et le rôle des stages sont cruciaux, afin d'endiguer la baisse du la baisse du nombre de médecins généralistes dans ces territoires. En effet, leur nombre a diminué de 10 % en dix ans selon l'ordre des médecins. Les CHU demeurent les acteurs centraux de la formation médicale pratique, mais ils valorisent sans doute trop une médecine hospitalière hyperspécialisée, au détriment de la médecine générale. Il faut non seulement renforcer la formation des étudiants à cette médecine, qui permet de prendre en compte le malade dans sa globalité familiale, sociale, culturelle et environnementale, ce que les CHU ne permettent pas, mais aussi inciter les étudiants à redécouvrir les pratiques spécifiques aux territoires ruraux, qui peuvent répondre à leurs attentes, notamment dans les hôpitaux locaux. À Buis-les-Baronnies dans la Drôme, une initiative intéressante a été mise en place : l'accueil des stagiaires par des médecins généralistes ayant reçu une formation spécifique de maître de stage s'est déroulé en lien avec l'hôpital local de la commune, hôpital qui loge à titre gracieux les stagiaires dont il attend en retour retour qu'ils accompagnent leur maître de stage lorsque celui-ci se rend dans l'établissement pour y suivre ses patients. Toutefois, cette organisation rencontre des obstacles, car il est encore difficile de faire reconnaître aux doyens des facultés et à leur département de médecine générale que les hôpitaux locaux puissent devenir des terrains de stage « validant Peut-être faudrait-il assouplir ces règles car, au-delà de cette initiative, les hôpitaux locaux peuvent jouer un rôle essentiel qu'il convient de développer pour lutter contre les déserts médicaux. Madame la ministre, pouvez-vous me faire part de votre avis sur la place que le Gouvernement souhaite donner aux hôpitaux locaux dans le cadre des études de médecine ? Comment comptez-vous aborder le problème du manque d'incitation des futurs médecins à s'installer dans les zones sous-denses,

les étudiants travaillent régulièrement 90 heures par semaine. L'ordre national des médecins parle d'ailleurs de burn-out à un stade d'évolution sévère pour près de deux internes sur trois. Un sur cinq développerait même des tendances suicidaires. Les risques psychosociaux auxquels ces jeunes sont confrontés s'expliquent aussi par les pressions qu'ils subissent lorsqu'ils tentent de revendiquer leurs droits. C'est donc à l'État de protéger ces apprentis médecins.

À l'image de ce qui se pratique en Grande-Bretagne pour les internes ou en France pour les praticiens hospitaliers, la réforme doit prévoir des dispositifs qui régulent les heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures de temps médical hebdomadaire. En d'autres termes, il est préférable de rémunérer ou de faire récupérer des heures supplémentaires au-delà des 48 heures de travail hebdomadaire, afin d'inciter les services à recruter de vrais médecins,

à rappeler que les internes sont à la fois des étudiants de troisième cycle inscrits à l'université et des agents publics affectés dans un CHU de rattachement, et rémunérés par ce dernier. En tant qu'agents publics, ceux-ci sont régis par un statut inscrit dans le code de la santé publique, qui prévoit des mesures relatives à leurs droits et à leurs obligations. Les dispositions qui leur sont applicables en matière de temps de travail sont donc adaptées à la spécificité de leur situation. Généralement, leur temps de travail est comptabilisé en demi-journées. Avant 2015, leurs obligations étaient fixées à onze demi-journées par semaine.

participation à la permanence des soins de ne pas voir leur temps de formation de jour et en stage réduit. Cette possibilité est actuellement étudiée par les services de mon ministère. Les garanties et conditions qui seraient susceptibles de l'encadrer sont particulièrement importantes en raison de la sensibilité que nous accordons tous aux questions relatives à la qualité de vie au travail. Je suis personnellement très attentive à l'évolution des discussions avec les internes.

mais surtout de l'inefficacité des différentes politiques et actions mises en place depuis deux décennies. C'est ce constat accablant que la commission du développement durable du Sénat faisait déjà en 2013, ... Eh oui ! ... dans un rapport de notre collègue Hervé Maurey. causes de ces déserts médicaux, le rapport apportait des réponses pragmatiques dans l'intérêt des territoires et de leurs habitants. Certaines visaient justement à faire évoluer les études de médecine, sans grand résultat jusqu'à présent. Et la désertification médicale est toujours aussi prégnante dans nos campagnes ! Madame la ministre, comment redonner vie à notre ruralité qui refuse de mourir ? Nous savons bien que la réforme des études de médecine ne produira pas d'effets avant une dizaine d'années. Il est donc nécessaire de prendre dès maintenant des mesures transitoires d'urgence, comme le préconise le professeur Patrice Diot, doyen de la faculté de Tours. C'est dans cet esprit que celui-ci devrait prochainement expérimenter la création d'un statut

de droits sociaux, comme ceux des assistants d'hôpitaux, par exemple. Madame la ministre, je souhaiterais connaître votre sentiment sur cette initiative, dernière chance d'obtenir une réponse concrète à une situation devenue dramatique ! Très bien ! La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je vais m'efforcer d'être brève. L'augmentation du national ne permet pas de répartir la hausse des étudiants de façon égale sur le territoire. Il y a davantage de médecins formés mais, en même temps, le rapport de la Cour des comptes

par exemple. Pourtant, avec ses 281 médecins pour 100 000 habitants en 2016, contre 421 en moyenne au niveau national, la région Centre-Val de Loire fait figure de désert médical. Malgré la hausse générale du, il reste donc de fortes inégalités territoriales. Le nouveau volet du pacte territoire-santé a permis de développer les stages des futurs médecins en cabinet de médecine générale et dans plusieurs spécialités médicales. Or aucune obligation n'existe sur la localisation de ces stages, notamment en zone peu dense. Madame la ministre, je souhaiterais que se développe le statut du médecin adjoint, expérimenté avec succès en Eure-et-Loir.

Mme la ministre. Madame la sénatrice, vous me parlez des stages en zone sous-dense. Comme je l'ai dit, nous essayons de développer de façon très proactive les stages en zone sous-dense en favorisant l'émergence de maîtres de stage notamment dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais aussi dans les cabinets

Nous avons impérativement besoin de diversifier l'offre de stage. La proposition que vous faites est déjà mise en oeuvre : les ARS sélectionnent les offres de stages avec les doyens. Nous les encourageons et essayons de faire en sorte qu'un

alors que le Président de la République a visité le CHU de Rouen ce matin, notre pays fait face à une modification certaine de la démographie de manière générale, et de la démographie médicale en particulier. Un plan pour renforcer l'accès territorial aux soins a été annoncé. Je félicite le Gouvernement d'avoir pris en compte la réalité de la situation. Comme vous le savez, il faut dix ans pour faire un médecin. Les études sont longues, le métier difficile. Si, en plus, on dit à des jeunes gens qui veulent choisir les études médicales qu'à la fin ils se retrouveront face à des mesures coercitives, j'ai peur qu'on ne les décourage encore bien davantage. La question du est sur la table depuis quelques années, comme si l'ouvrir largement était une panacée. Nous savons bien que l'université comme l'hôpital ne sont pas en mesure d'accueillir aujourd'hui massivement plus d'étudiants. Ces études sont trop concentrées sur l'hôpital. Si les étudiants apprennent leur art en milieu hospitalier, ils n'ont bien souvent aucune idée de ce qu'ils verront et feront en ville. Néanmoins, je ne peux aborder la question de l'hôpital sans évoquer l'ensemble du personnel hospitalier, qu'il soit soignant, technique ou administratif. Je voudrais lui rendre hommage en ces temps où l'on parle beaucoup de souffrance au travail. Il apparaît presque ironique que la communauté médicale, qui est au premier rang de la prise en charge de cette souffrance, compte parmi les professions les plus touchées par le burn-out. Une ouverture sur la médecine de ville, des stages dès le deuxième cycle, serait nécessaire pour permettre aux futurs médecins de mieux se préparer. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles sont vos intentions dans le décloisonnement ville-hôpital, et ce dès la formation des soignants ?

sanitaire : celui-ci a été lancé et sera opérationnel dès le mois de septembre prochain pour les 45 000 étudiants en santé, dont les 8 700 nouveaux médecins. Cet exercice sanitaire va permettre aux jeunes médecins de faire de la prévention et de l'éducation à la santé dans différents endroits, notamment les collèges ou les lycées, mais surtout

et fondé sur les matières scientifiques. Ne peut-on pas diversifier le profil des étudiants qui intègrent les études de médecine ? Nous avons un travail à engager sur les besoins en termes de démographie médicale en 2035-2040, parce qu'un certain nombre de métiers vont évoluer, notamment tous les métiers de l'imagerie qui vont se transformer

Faisant le constat que l'on forme davantage de futurs praticiens hospitaliers que des médecins de ville- je rappelle que dès la troisième année de médecine les étudiants sont en quasi-permanence à l'hôpital nous proposions notamment de modifier les critères de sélection pour favoriser une plus grande mixité sociale et géographique, de diversifier l'enseignement en introduisant des matières favorisant l'installation en ambulatoire, que ce soit la gestion, la communication ou l'économie de la santé, de la santé, et de rendre réellement obligatoire la réalisation d'un stage en médecine générale permettant de valider le deuxième cycle. Ce rapport préconisait également de réformer les épreuves classantes nationales. Ce système où des QCM déterminent l'avenir des étudiants en termes de spécialisation et d'affectation géographique, sans prendre en compte leurs résultats aux examens antérieurs ou le bilan de leurs stages doit incontestablement être revu. J'ajoute, mais vous le savez, madame la ministre, qu'un écart d'un dixième de point modifie parfois de plusieurs milliers de places le classement et, par là même, l'avenir des étudiants. J'aimerais donc savoir si vous comptez revoir ce système. De même, si vous réduisez la présence des étudiants externes et internes dans les hôpitaux pour favoriser une meilleure connaissance de la médecine libérale, ce qui me semble souhaitable, comment fonctionneront les hôpitaux,

nouveaux lieux de stage pour les internes en zone sous-dense dans le plan d'accès aux soins, ... Très bien ! ... en plus des 350 postes de maître de stage qui vont être financés en zone sous-dense dès cette année.

Or ceux-ci doivent, selon moi, rester au centre du système de santé. Il n'est pas concevable de compenser le manque de médecins par le recours à des infirmiers ou des infirmières, qui sont, certes, leurs collaborateurs les plus précieux, indispensables pour suivre les patients et donner les alertes, mais qui ne sauraient en aucun cas se substituer à eux.

mais réservée aux facultés établies sur des territoires évoluant en déserts médicaux, en tenant compte, aussi, de l'âge des médecins ? Cette augmentation de 10 % serait fléchée vers des étudiants qui souhaiteraient se mettre au service d'un territoire dans le besoin.

qui permet la régionalisation. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour deux minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la réforme du troisième cycle des études de médecine, initiée à la suite du rapport des professeurs François Couraud avait pour objectif de résoudre les problèmes posés par l'internat : absence d'interdisciplinarité, insuffisance de lien entre les différents stages effectués par les internes ou encore manque de régulation des places en diplôme d'études spécialisées complémentaires, Mise en oeuvre à la rentrée 2017, la réforme restructure totalement l'organisation du troisième cycle. Elle a ainsi supprimé les DESC qui permettaient aux médecins de revendiquer une double spécialisation, double spécialisation, ce qui n'est pas sans soulever quelques difficultés. Je pense tout particulièrement à la médecine d'urgence. Avant la réforme, un interne en

Aujourd'hui, ces passerelles ne sont plus possibles, la médecine d'urgence étant devenue une spécialité à part entière. Si je peux comprendre que le système précédent ne permettait pas de savoir exactement combien d'internes en médecine générale exerceraient bien la médecine générale en fin d'études, et ainsi de répondre au mieux à la demande de soins sur le territoire, il ne me semble pas raisonnable de penser qu'un médecin urgentiste exercera ce métier toute sa vie. Selon une étude, la carrière de médecin urgentiste durerait en moyenne sept ans Madame la ministre, ne craignez-vous pas que les jeunes médecins qui souhaitent travailler seulement quelques années aux urgences ne finissent par choisir une autre spécialité ? Ne craignez-vous pas de perdre ainsi des vocations ? Mme la ministre. Monsieur le sénateur, vous posez une excellente question. Il se trouve que le DESC de médecine d'urgence a été réclamé

à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, le service sanitaire a été conçu pour atteindre deux objectifs principaux. Le premier, c'est que nos étudiants intègrent complètement la prévention et l'éducation à la santé dans leur pratique.

un suivi de ce service sanitaire avant son déploiement sur l'ensemble des professionnels de santé. Aujourd'hui, il ne concerne que 6 professions de santé et 48 000 étudiants, mais nous devrions aller jusqu'à 50 000 étudiants

Comme vous le savez, de par leur géographie, leur isolement et leur situation démographique, les outre-mer en général, et plus particulièrement la Guyane, sont extrêmement touchés par la désertification médicale. La Guyane est l'un des départements français le moins favorisé pour les indicateurs de santé, ce qui lui confère une situation sanitaire fort préoccupante. En effet, le sous-développement général en matière d'infrastructures et de professionnels de santé place le territoire en situation de crise chronique. Si des efforts sont faits, ils ne suffisent pas à rattraper le retard accumulé dans un contexte de forte croissance démographique. Pour ces raisons, les études de médecine constituent un véritable enjeu de développement pour la Guyane. Nous disposons bien d'une université de plein exercice depuis le 1 janvier 2015, mais seule la première année commune aux études de santé- PACES -y est dispensée, avec, toujours, un rattachement à l'université des Antilles. d'enseignants est faible. Les cours se déroulent en visioconférence ou sur supports vidéo. Force est de constater que les conditions actuelles de formation ne permettent pas de préparer davantage d'étudiants en PACES et, donc, de futurs médecins. Pour rappel, la Guyane ne disposait que de douze places en médecine pour 2018. Pourtant, et vous en conviendrez, le développement économique et social passe aussi bien par l'accompagnement vers la réussite de la jeunesse que par un accès aux soins de qualité. Dans ce contexte, madame la ministre, comment faire des études de médecine un moyen d'action pour lutter plus efficacement contre la désertification médicale outre-mer ? S'agissant de la Guyane, le Gouvernement est-il prêt à étudier sérieusement l'opportunité de créer une faculté de médecine de plein exercice, afin d'ouvrir le et de permettre à nos étudiants de poursuivre leur deuxième et troisième cycles sur le territoire guyanais ? La parole est à Mme la ministre.

nous avons souhaité un renforcement des liens avec les services et les facultés des Antilles et nous allons poursuivre nos encouragements en ce sens. Nous allons également favoriser l'accueil en stage d'étudiants de deuxième et de troisième cycle,

Il s'agit d'une année inhumaine, qui a des conséquences terribles sur la santé des étudiants et des étudiantes. Notons que 70 % d'entre eux souffrent de symptômes dépressifs et que la consommation d'anxiolytiques ou de drogues est très élevée. ou de drogues est très élevée. Sous la pression de cette hypersélection, les étudiants et les étudiantes achètent très majoritairement les services d'officines privées, pour des montants élevés- de 4 000 à 5 000 euros. C'est une forme de sélection sociale, qui exclut encore plus les étudiants aux revenus les plus modestes.

Cet apparent paradoxe m'oblige donc à vous demander, madame la ministre, si la forme d'organisation de la PACES- son mode de sélection, le recours à l'offre privée, le -n'est pas une anticipation de ce que seront les autres années universitaires après la mise en oeuvre de la loi ORE. La

Toutes les possibilités sont sur la table. Je ne veux pas m'engager dès lors que les consultations ne font que débuter. Nous nous sommes donné jusqu'à la fin de l'année pour élaborer une réforme globale

de notre population. Madame la ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que le présent débat a été inscrit par la conférence des présidents dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe du RDSE, soit

Il reviendra à la conférence des présidents d'inscrire éventuellement la suite de ce débat à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Je n'ai été saisie d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents. Elles sont donc adoptées.